Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des lois a été publiée.

aux droits des femmes -chère Annick Billon -, madame la rapporteur -chère Marie Mercier -, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le projet de loi dont nous allons débattre aujourd'hui, qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, est le fruit d'un long travail engagé bien avant l'élection du Président de la République. En effet, lors de sa campagne, il avait pris l'engagement de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale de son quinquennat. Cette promesse a été tenue dès le discours prononcé le 25 novembre dernier intronisant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles subies quotidiennement par des millions de femmes comme première priorité de cette grande cause quinquennale. Ce projet de loi constitue une réponse, que je crois efficace et concrète, aux attentes exprimées cet automne, lors du tour de France de l'égalité, la plus grande consultation citoyenne jamais organisée par un gouvernement, avec plus de 830 ateliers sur l'ensemble du territoire. Aussi, je voudrais de nouveau devant vous remercier les 55 000 participantes et participants qui ont contribué à enrichir le projet du Gouvernement, faisant de ce texte la première grande loi citoyenne du quinquennat. Malgré les avancées enregistrées au cours des deux dernières décennies, les statistiques restent désespérément stables d'année en année. Pire encore, en dépit du récent mouvement que l'on a appelé de libération de la parole ou de libération de l'écoute, la réalité et l'ampleur de ces violences sont certainement toujours sous-estimées, notamment parmi les plus jeunes d'entre nous. Pour des enfants, parler des violences dont ils sont victimes et être assurés qu'on les croira lorsqu'ils les dénoncent reste bien trop souvent insurmontable. Je note par ailleurs que l'absence de données fiables relatives aux violences sexuelles commises sur les hommes montre bien le poids du tabou ou du déni qui contribue à rendre ces actes indicibles, et donc invisibles. Le temps de l'omerta est révolu et il est de notre responsabilité collective de faire reculer toutes ces formes de violence. Je sais que toutes et tous, ici, vous partagez cette conviction, et c'est avec détermination et humilité que le Gouvernement présente aujourd'hui devant la Haute Assemblée ce projet de loi. Je ne peux pas ne pas évoquer ici, au Sénat, devant vous, la mémoire de Jean-Claude Boulard, qui fut sénateur, et qui nous a quittés voilà quelques semaines. Il m'a fait entrer en politique fait qu'il avait, chevillée au corps, la conviction de l'utilité du bicamérisme, puisqu'il disait, permettez-moi de le citer : « Lorsque j'écris un texte, je le fais toujours lire deux fois par deux groupes différents de personnes, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que seul. » Merci pour lui ! Je tiens à saluer la qualité de vos travaux sur ce sujet sensible ; elle illustre notre souci commun de défendre l'intérêt des plus vulnérables. Je crois que le point commun de vos travaux et des nôtres, c'est qu'ils sont fondés sur le même constat : trop peu d'agresseurs sont poursuivis et sanctionnés. Alors que 10 % des victimes de violences sexuelles portent plainte, il y a urgence à agir pour renforcer leur protection et garantir l'exercice de leurs droits. Chacun sait ici l'importance de ces objectifs qui nous réunissent : mieux prévenir les violences, bien sûr, mieux protéger les victimes et, en ce qui concerne ce projet de loi, mieux sanctionner les agresseurs. Nous avons naturellement des divergences sur les moyens de répondre à ces exigences, mais je ne doute pas une seconde de votre engagement pour faire en sorte que nous parvenions ensemble à un texte qui soit le plus efficace possible. Je voudrais d'ailleurs souligner que nos propositions présentent certaines similitudes. C'est le cas, par exemple, sur l'allongement des délais de prescription à trente ans, sur l'extension de la surqualification d'inceste aux victimes majeures, sur l'aggravation des sanctions encourues pour l'atteinte sexuelle. Il m'apparaît que, au-delà de certaines divergences d'opinion légitimes, il y a des dispositions sur lesquelles nous pourrons nous rejoindre au cours des débats. Le texte que vous allez examiner, qui a été amélioré en première lecture par l'Assemblée nationale, est, je le crois, un texte fort fort permettant de mieux protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment parce qu'il apporte des réponses juridiques fortes à des réalités qui, trop longtemps, sont restées dans les angles morts des politiques publiques. Je pense ici à la disposition visant à sanctionner le harcèlement dit « de rue Lors de sa campagne, le Président de la République s'était engagé sur ce sujet, répondant à l'attente très forte exprimée par nos concitoyens et, bien sûr, par nos concitoyennes. Je rappelle qu'une étude très très récente de l'IFOP nous a appris que 8 jeunes femmes sur 10 ont peur de sortir seules dans la rue le soir, en France, en 2018 ... Et je me permets de vous avouer ici mon étonnement de constater que cette mesure tant attendue ne fait pas consensus, semble ne pas faire consensus dans cet hémicycle. En effet, au terme des débats qui ont déjà eu lieu, il semblerait que vous ne partagiez pas l'avis du Gouvernement sur l'importance de sanctionner ces agissements subis chaque jour par des millions de personnes, quels que soient leur genre, leur orientation sexuelle ou leur identité. Vous proposez de faire du harcèlement de rue un délit. Je m'interroge sur ce choix, car je crois, mais nous en débattrons, que cela n'est pas applicable. J'ai en tête l'échec de la loi belge, qui a bien montré les limites de ce type de dispositif, avec seulement trois plaintes déposées, toutes classées sans suite. Ne refaisons pas les mêmes erreurs et soyons pragmatiques pour être efficaces. C'est pour cette raison que le Gouvernement a choisi de proposer une nouvelle infraction, celle de l'outrage sexiste, qui pourra être sanctionnée par une contravention en flagrance par les 10 000 policiers de la sécurité du quotidien.

les relations entre les femmes et les hommes peuvent s'établir en confiance, doivent s'établir en confiance ; il est de notre responsabilité de permettre le respect mutuel que chacun mérite, femme ou homme, et ce partout dans la société, à commencer par l'espace public, où chacune et chacun doit pouvoir être libre d'aller et de venir sans crainte. Ce respect mutuel doit aussi être garanti sur Internet. C'est pourquoi nous proposons de mettre fin à ce sentiment d'impunité que peuvent ressentir des agresseurs en ligne se cachant derrière l'écran et derrière l'anonymat pour donner libre cours à la misogynie. Les jeunes sont massivement touchés par ces violences en ligne, mais pas uniquement eux : plus de trois quarts des adolescents ne savent pas comment réagir face au cybersexisme -76 %, selon l'étude du Centre Hubertine Auclert. Auclert. Il nous faut répondre de manière forte à ce phénomène, qui est aussi destructeur dans le monde virtuel que dans le monde réel. Toutes ces formes de violence qui se développent dangereusement doivent être sanctionnées. Tel est l'objet de l'article 3 du projet de loi, adapter notre arsenal juridique à ces nouvelles possibilités qu'Internet offre aux agresseurs. Cet article vise particulièrement les « raids numériques », c'est-à-dire la publication par plusieurs personnes différentes de propos sexistes et violents, proférés à l'encontre d'une même cible. Une telle forme de violence n'entre pas aujourd'hui dans les définitions actuelles du harcèlement, qui est constitué par la répétition de faits par une même personne. L'article 3 du projet de loi va donc élargir la définition du harcèlement pour y intégrer cette notion de concertation et punir désormais ces raids numériques qui, jusqu'à présent, contribuaient à donner le sentiment qu'Internet pouvait être une zone de non-droit, ce que nous ne pouvons pas Nous voulons donc envoyer un message clair aux harceleurs en ligne, à ceux qui incitent ou prennent part à ces opérations de déferlement de haine en ligne, en disant qu'elles seront désormais clairement punies par la loi. À l'occasion de la première lecture de ce projet de loi au Sénat, le Gouvernement souhaite réaffirmer sa volonté d'adapter la répression aux nouvelles formes que les violences sexuelles et sexistes peuvent prendre.

ou d'abuser de l'état d'ivresse dans lequel elle se trouve. De tels agissements constitueront désormais une circonstance aggravante des infractions sexuelles. La limite, c'est le consentement, et il n'est pas tolérable en France, en 2018, que cette notion de consentement ne soit pas universelle. C'est pourquoi nous proposons que le fait d'administrer, à l'insu de la victime, une substance qui vise à altérer son discernement

comble un vide juridique, encore une fois. Elle vise à sanctionner la captation d'images, dites « impudiques », à l'insu de la personne. C'est un phénomène trop répandu, en hausse, notamment dans les transports en commun. Ce sujet nous est remonté au cours des échanges que nous avons continué à mener depuis la présentation du projet de loi, et qui sont venus enrichir notre réflexion. Ces faits de voyeurisme ne sont pas réprimés aujourd'hui. Comme le cyberharcèlement, comme le harcèlement de rue, ils n'entrent pas aujourd'hui dans les infractions existantes. Nous proposons donc de créer un nouveau délit, puni de un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

considérable sur la vie des victimes, de l'angoisse éprouvée quotidiennement dans une rue, parfois déserte, sur le chemin du travail, jusqu'aux psychotraumas les plus sévères. On sait aujourd'hui que les viols causent des traumatismes similaires à ceux qui Les conséquences des violences sexuelles sur la santé physique et mentale sont d'autant plus graves que les victimes sont jeunes. C'est la raison pour laquelle, comme l'évoquera, je pense, ma collègue garde des sceaux, deux des quatre dispositions de notre projet de loi concernent les infractions sexuelles commises sur mineur. L'allongement à trente ans du délai de prescription applicable aux crimes commis à l'encontre des mineurs est un rouage essentiel d'une meilleure protection des plus vulnérables. Votre assemblée semble partager cette conviction, ce dont je ne peux que me réjouir. Je sais que la dernière réforme de la prescription est récente, avec la loi Fenech-Tourret de 2017, mais l'évolution que nous proposons est nécessaire, je le crois, pour mieux prendre en compte la difficulté des victimes à révéler les faits, notamment en raison du phénomène d'amnésie traumatique, mais aussi à cause de la difficulté de verbaliser et de judiciariser ces faits. Je suis donc heureuse que nous fassions le même constat, conformément aux recommandations de la mission de consensus menée l'an dernier, sous la direction de Flavie Flament et de Jacques Calmettes, sur l'initiative de ma prédécesseure, la sénatrice Laurence Rossignol, que je salue. Nous souhaitons cependant rétablir par voie d'amendement l'allongement du délai de prescription applicable à l'ensemble des crimes sur mineurs, dont le meurtre, par souci de cohérence et pour faciliter l'exercice de poursuites judiciaires de nombreuses années après les faits. Nous vous proposons même d'améliorer encore cette disposition afin d'éviter l'impunité des personnes qui commettent, pendant de très longues périodes, ces crimes sur des mineurs, de façon répétée. pour éviter que les faits les plus anciens ne soient prescrits, nous proposons que la commission de nouveaux crimes interrompe la prescription des crimes les plus anciens. Il peut s'agir, par exemple, de faits d'inceste commis sur plusieurs générations. Notre droit, je le crois, doit reconnaître l'exceptionnelle gravité des crimes qui sont commis sur les mineurs. C'est pourquoi non seulement nous créons des conditions plus favorables à la libération de la parole des victimes, mais encore nous renforçons cet arsenal juridique. cet arsenal juridique. Nous souhaitons donc renforcer la protection des mineurs et mieux sanctionner leurs agresseurs. Vous connaissez la position du Gouvernement à l'égard des modifications apportées à l'article 2, dont la rédaction avait été précisée et améliorée par l'Assemblée nationale, et dont l'objectif unique est bien d'éviter au maximum les acquittements des auteurs d'infractions sexuelles. À cet égard, je voudrais d'abord souligner l'importance du maintien du caractère interprétatif de la première disposition de l'article 2, qui permet d'échapper à la non-rétroactivité de la loi pénale. Ainsi, le juge pourra s'en saisir dès la promulgation de la loi pour toute affaire, y compris en cours, ce qui peut concerner des millions de victimes du fait de l'allongement des délais de prescription. C'est le caractère interprétatif cela. Je souhaite rappeler que nous nous rejoignons, me semble-t-il, mais les débats nous le dirons, sur la nécessité d'affirmer qu'un mineur en dessous d'un certain âge n'est jamais consentant à un acte sexuel avec un majeur. Il s'agit là, je le pense, d'un véritable enjeu de civilisation. Nous en sommes toutes et tous convaincus. Pour autant, vous connaissez nos réserves sur votre proposition d'instaurer une présomption de contrainte, qui est une option présentant, de notre point de vue, des risques d'inconstitutionnalité. C'est ce que nous a démontré le Conseil d'État. Enfin, nous partageons votre souci d'améliorer les modalités de la mise en oeuvre de la question subsidiaire. Comme l'a rappelé le président de votre commission des lois, Philippe Bas, le Sénat prend le temps du travail, de la réflexion, et, même si ce point semble être un détail, son importance juridique est essentielle. J'en viens à l'un des points importants de notre discussion. Depuis plusieurs mois, un certain nombre d'associations de protection de l'enfance, mais aussi de professionnels du droit, de la santé, ou de travailleurs sociaux nous interpellent et échangent avec nous sur les risques que pourrait présenter la disposition relative à l'augmentation des peines encourues pour atteinte sexuelle

Je suis heureuse de vous annoncer que, fidèles à l'esprit de concertation qui nous a animés tout au long de l'élaboration de notre projet de loi, nous avons écouté et entendu ces inquiétudes pour finalement prendre en compte les réserves exprimées, y compris par les sénatrices et les sénateurs. Aussi, parce qu'il ne veut pas brouiller le message que porte ce texte, le Gouvernement a fait le choix de ne pas réintroduire cette disposition lors de la première lecture au Sénat, et nous ne le ferons pas non plus à l'occasion des prochaines discussions de ce texte. Nous suivons donc les avis que vous avez souhaité rendre et les dispositions que vous avez souhaité prendre en commission des lois du Sénat. Ce choix, je le crois, c'est celui de la cohérence et de la raison. Nous voulons toutes et tous mieux protéger tous les enfants, et nous ne voulons pas prendre le risque, si infime soit-il, d'envoyer un mauvais message aux agresseurs ou d'exposer ne serait-ce qu'une seule victime à la possibilité d'une déqualification du crime qu'elle aurait subi. Nous pensions que cette disposition était utile ; après vous avoir écoutés, nous avons donc

dernier, une figure du combat pour les droits des femmes est entrée au Panthéon, après être entrée dans l'histoire de notre pays comme dans le coeur des Françaises et des Français. Lors de nos débats, nous essaierons de nous montrer dignes de l'héritage que nous a légué Simone Veil, particulièrement à nous, les à nous, les femmes. Simone Veil disait souvent qu'il suffit d'écouter les femmes. C'est dans cet état d'esprit, à l'écoute, que nous entendons nous placer lors des débats que nous aurons ensemble. Je crois que nous pourrons alors collectivement être fiers d'agir en faveur des droits des femmes, à l'heure où, insidieusement, ils sont remis en cause, partout dans le monde,

de notre ambition commune de mieux prévenir, de mieux sanctionner toutes ces formes de violence qui procèdent toujours de la volonté de soumettre, de détruire l'autre en instrumentalisant son corps, qu'il s'agisse d'une femme, d'un enfant, et même d'un homme. Faisons en sorte aujourd'hui, partout, à chaque instant, que toutes et tous soient mieux protégés, que les agresseurs soient davantage condamnés et que le signal envoyé par la République française soit extrêmement clair à cet égard : nous nous tenons avec les victimes, pour la condamnation des agresseurs. Au-delà des clivages, il nous appartient à toutes et à tous d'en faire un moment marquant d'une avancée de notre droit et de l'Histoire. La parole Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois - cher Philippe Bas -, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes - chère Annick Billon -, madame la rapporteur

de mobiliser l'ensemble de nos moyens pour que, sur le sujet des violences faites aux femmes et aux enfants, désormais « la honte change de camp Le texte que nous portons, dans sa version enrichie par les apports des députés qui l'ont adoptée le 16 mai dernier, doit permettre d'améliorer très significativement notre arsenal législatif répressif concernant les violences faites aux femmes et aux enfants.

l'article 1 allonge le délai de prescription de l'action publique des crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs, en le faisant passer de vingt ans à trente ans ans à compter de la majorité de ces derniers. Cette modification est apparue indispensable afin de laisser davantage de temps aux victimes pour porter plainte et faciliter la répression de ces actes, notamment lorsqu'ils sont incestueux. Cet allongement de la prescription, il faut le souligner, est tout d'abord cohérent avec l'augmentation générale des délais de prescription, telle qu'elle a été opérée par la loi du 27 février 2017.

donc plus long que celui de la prescription de droit commun. Il n'est donc pas absurde de rétablir une différence temporelle qui préexistait entre la prescription des crimes de droit commun et celle des crimes sexuels sur mineurs. Cet allongement est ensuite essentiel pour donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits, en prenant notamment en compte les mécanismes de la mémoire traumatique, et éviter ainsi l'impunité de leurs auteurs. Le délai de trente ans commençant à courir à compter de la majorité de la victime, il permettra ainsi à cette dernière de révéler les faits jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de quarante-huit ans, au lieu de trente-huit ans actuellement.

que pour les crimes « touchant l'ensemble de la communauté internationale », ce qui n'est pas le cas des crimes commis à l'encontre des mineurs, en dépit de leur extrême gravité.

afin de répondre à l'incompréhension suscitée par des affaires judiciaires récentes dans lesquelles des fillettes de onze ans ont, du moins dans un premier temps, été considérées comme ayant consenti à des rapports sexuels avec des hommes majeurs. sexuels avec des hommes majeurs. Tout d'abord, en matière de viol et d'agression sexuelle, l'article 2, tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale, complète l'article 222-22-1 du code pénal afin de préciser : « : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale [ ...] ou la surprise [ ...] sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes Ensuite, en matière d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, cet article double les peines encourues, à hauteur de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, lorsqu'un acte de pénétration sexuelle a été commis par le majeur.

la qualification d'atteinte sexuelle devra obligatoirement être posée par le président de la cour d'assises si l'existence de violences, contrainte, menace ou surprise est contestée.

ont reçu un avis défavorable du Gouvernement, tant pour des raisons constitutionnelles qu'en opportunité. Ils ont donc été rejetés par l'Assemblée nationale. Sur la question de l'âge, tout d'abord, il ne nous est pas paru possible de prévoir des règles spécifiques pour les mineurs de treize

Surtout, la fixation d'un seuil de treize ans donnerait, à tort, l'impression qu'une atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur plus âgé, notamment sur des mineurs de quatorze ans et quelques mois ou d'un peu moins de quinze ans, serait licite ou tolérable, ce qui n'est évidemment pas acceptable.

l'institution de présomptions légales en matière criminelle semble contraire aux exigences constitutionnelles de respect de la présomption d'innocence.

elles qui me paraissent directement inspirées des travaux menés par le Sénat dans la proposition de loi qui a été examinée et débattue au mois de mars dernier. Il en est ainsi de l'extension de la surqualification d'inceste aux victimes majeures, de l'aggravation de cinq à sept ans de la peine d'emprisonnement encourue en matière d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, ou encore de l'aggravation des peines d'emprisonnement de cinq pour le délit de non-assistance à personne en danger et de trois à cinq ans pour le délit de non-dénonciation de mauvais traitements, lorsque ces délits sont commis sur un mineur de quinze

améliorer notre législation en matière de lutte contre toute forme de harcèlement, qu'il soit commis sur internet ou dans la rue. Marlène Schiappa vous en a déjà présenté l'économie générale. ces éléments de présentation du projet de loi étant posés, je vous ferai maintenant part de quelques observations du Gouvernement sur le travail de la commission des lois du Sénat.

la particulière qualité du travail conduit par la commission des lois, qui s'explique notamment par l'intérêt que la Haute Assemblée porte depuis plusieurs années à la question des violences sexuelles commises sur les femmes et sur les enfants.

Cet intérêt résulte également des travaux accomplis par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Je souhaite donc ici vivement remercier votre rapporteur, Marie Mercier, et les membres de la délégation, du travail de longue haleine qu'ils réalisent sur ces sujets.

conduit à ce qu'il existe, sur de nombreux points, d'importantes convergences de vue et d'analyse entre le Sénat et le Gouvernement, concernant précisément les quatre mesures phares du projet de loi. Ainsi votre commission Ainsi votre commission est-elle favorable à une augmentation de vingt à trente ans de la prescription des crimes de nature violente ou sexuelle commis sur des mineurs, n'était une divergence minime concernant la liste de ces crimes, divergence qui, j'en suis persuadée, pourra être surmontée. De même, votre commission accepte, dans son principe et dans la quasi-intégralité de sa rédaction, la disposition interprétative précisant la notion de contrainte ou de surprise en cas d'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze Cela permettra- tel est bien son objectif -aux juridictions de retenir plus facilement et plus fréquemment les qualifications de viol et d'agression sexuelle. Par ailleurs, votre commission accepte l'évolution de la définition relative à l'élément de répétition des faits caractérisant le délit de harcèlement sexuel, ce qui permettra de sanctionner les harcèlements numériques commis par plusieurs internautes. votre commission accepte le principe de la création d'une infraction d'outrage sexiste pouvant être réprimée par la procédure de l'amende forfaitaire. Ces convergences de vue me semblent plus importantes que nos différences. La première divergence La première divergence concerne la question de la présomption de culpabilité. S'agissant des violences sexuelles commises sur des mineurs de quinze ans, votre commission propose, dans certains cas, la création d'une présomption de contrainte, donc de culpabilité. cela ne nous semble pas possible au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son avis, l'instauration d'une présomption en la matière serait très très difficilement compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, en dehors du champ contraventionnel, lorsque les faits peuvent raisonnablement induire la vraisemblance de l'imputabilité- c'est le cas, par exemple, des infractions au code de la route relevant de cette catégorie

d'une part, qu'elle ne revête pas de caractère irréfragable, d'autre part, qu'elle assure le respect des droits de la défense, c'est-à-dire qu'elle permette au mis en cause de rapporter la preuve contraire. Ces exigences seraient nécessairement d'autant plus fortes si une telle présomption devait être être instituée pour un crime. Au demeurant, toujours selon le Conseil d'État, la même présomption, s'agissant d'un crime, excéderait très certainement « les limites raisonnables » dans lesquelles la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales enserre les présomptions de droit ou de fait en matière pénale, compte tenu de la gravité de l'enjeu et de la difficulté pour le mis en cause de se défendre

Le Gouvernement n'y est pas favorable, estimant qu'une incrimination contraventionnelle permettra une répression plus rapide et plus efficace des faits. Par ailleurs, si cette contravention est créée par la loi, alors que cela relève en principe du décret, c'est parce qu'une loi nous semble, en tout état de cause, nécessaire. Elle est nécessaire pour établir des amendes forfaitaires minorées, celles-ci n'étant aujourd'hui possibles, aux termes de la loi, que pour les contraventions au code de la route. Elle l'est aussi pour prévoir la peine complémentaire de stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Plutôt que de procéder en deux temps et de modifier la loi pour prendre ensuite un décret, tout régler dans la loi a paru une solution plus efficace et plus opportune au regard de la dimension symbolique de l'incrimination.

La question était de savoir s'il convenait de porter de cinq à dix ans d'emprisonnement la peine encourue en cas d'atteintes sexuelles commises sur un mineur de quinze ans lorsque ces faits sont commis avec pénétration. Le Gouvernement estimait que cette aggravation, qui lui avait été proposée par le Conseil d'État dans son avis, était opportune et justifiée pour affirmer avec force l'interdiction absolue de toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de quinze ans, que cette relation constitue un viol ou qu'elle n'en constitue pas un. Cette aggravation venait ainsi compléter la définition interprétative facilitant l'établissement de la contrainte ou de la surprise qui caractérisent le viol. Pour

certaines associations, qui ont cru y déceler une possibilité accrue de correctionnalisation des crimes de viol en délits d'atteinte sexuelle. cette perception est erronée, le Gouvernement ayant exclusivement souhaité renforcer les sanctions relatives aux violences sexuelles commises sur les mineurs. Avec mes collègues Agnès Buzyn et Marlène Schiappa, nous avons pris le temps de recevoir ces associations pour échanger avec elles et leur expliquer la démarche voulue par le Gouvernement sur ce point. Ces échanges ont été très riches, très francs, sans doute même enrichissants de part et d'autre. Plusieurs des représentants de ces associations nous ont dit comprendre notre démarche, mais nous ont indiqué redouter que, à vouloir trop bien faire, notre projet perde en lisibilité auprès de leurs membres et des victimes qu'elles côtoient sur le terrain chaque jour. Or l'intention du Gouvernement n'est certainement pas de susciter l'incompréhension de nos concitoyens ; elle est de travailler conjointement avec l'ensemble des forces de la société civile à l'affirmation et à la mise en place d'une dynamique sociétale globale de renforcement de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Pour atteindre ce but, nous devons être unis. Il nous est donc apparu nécessaire, à ma collègue Marlène Schiappa et à moi-même, de rassurer sur ce point le milieu associatif. Votre commission des lois a proposé de supprimer cette disposition relative à l'atteinte sexuelle avec pénétration Le Gouvernement, à la réflexion, accepte cette suppression, car il estime essentiel que ce projet de loi ne soit pas mal compris et mal perçu par ceux-là mêmes dont le rôle est fondamental dans la lutte contre les violences sexuelles commises sur les mineurs. Par ailleurs, l'Assemblée nationale, reprenant du reste une proposition initialement formulée par le Sénat, a porté de façon générale de cinq à sept ans d'emprisonnement la peine prévue en cas d'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, qu'il y ait ou non pénétration. Dans la logique d'instauration d'un répressif que j'évoquais précédemment, une telle aggravation peut paraître suffisante. Pour ces raisons, le Gouvernement ne proposera pas de revenir sur cette suppression. Il n'a donc déposé J'ajoute, pour finir, que le Gouvernement a déposé trois amendements

en permettant de prendre en compte la situation des personnes commettant de façon répétée des violences sur les mineurs. Il prévoit ainsi que la commission d'un nouveau crime avant la prescription d'un précédent crime interrompra cette prescription et permettra ainsi de poursuivre et condamner la personne pour l'ensemble de ses actes. Les deux amendements suivants complètent le projet de loi par deux dispositions

Ces dispositions ne figuraient pas dans le projet de loi initial, car il avait été alors décidé que celui-ci ne traiterait que des quatre réformes annoncées par le Président de la République dans son discours du mois de novembre 2017, à savoir la prescription, le viol sur mineur, le harcèlement sexuel sur internet et l'outrage sexiste. La première lecture à l'Assemblée nationale s'est principalement focalisée sur ces quatre questions. Considérant que l'examen du texte devant le Sénat constitue une étape importante et précieuse de la discussion parlementaire,

vise à renforcer les moyens juridiques à disposition de l'autorité judiciaire pour lui permettre de faire respecter au quotidien les droits des femmes et des enfants en mettant fin au sentiment d'impunité des auteurs de violences sexuelles et sexistes. Ce texte constitue une avancée majeure pour atteindre ce but que nous nous sommes collectivement fixé.

Madame la présidente, madame le garde des sceaux, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, que celles-ci concernent les femmes ou les hommes, les mineurs ou les majeurs, est un sujet sociétal gigantesque qui nous tient particulièrement à coeur. Ce sujet Ce sujet n'est pas nouveau. Nous en avons déjà débattu, notamment dans le cadre du groupe de travail pluraliste de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, qui a étroitement associé la délégation aux droits des femmes Le sujet a également été longuement évoqué lors de l'examen de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, présentée par le président de la commission des lois et adoptée le 27 mars dernier à la quasi-unanimité.

il propose à cette fin d'allonger certains délais de prescription, de mieux réprimer les viols commis à l'encontre des mineurs, ou encore de mieux réprimer les faits de harcèlement sexuel ou moral, notamment lorsqu'ils sont commis sur internet. La commission des lois a tenu à aborder ce texte dans un esprit constructif. Nous partageons tous les mêmes objectifs que le Gouvernement. Il est indispensable de continuer le combat contre les violences sexuelles et sexistes, violences qui touchent en majorité les femmes, mais aussi et trop souvent les mineurs, filles comme garçons. Comme le Gouvernement, nous considérons qu'il est essentiel de lutter contre les comportements sexistes dont sont victimes les femmes dans l'espace public. Ces comportements anciens sont trop souvent tolérés, banalisés, voire intégrés par les femmes elles-mêmes, qui ont tendance à adapter leurs comportements et leurs déplacements en fonction de ce risque. Comme le Gouvernement, nous considérons que les violences sur internet ne sont pas virtuelles. Bien que peu médiatisées, elles n'en restent pas moins réelles, avec des conséquences psychiques et physiques tout aussi dramatiques. Si la commission des lois a partagé sans réserve les objectifs du projet de loi, elle a néanmoins eu à coeur d'améliorer l'efficacité de certaines mesures et, évidemment, de reprendre l'ensemble des dispositions que le Sénat avait adoptées le 27 mars dernier lors du vote de la proposition de loi de Philippe Bas. Certaines de ses dispositions avaient déjà été reprises à l'Assemblée nationale. Ainsi, l'article 2 du projet de loi a été modifié afin d'étendre la surqualification pénale de l'inceste aux viols et autres agressions sexuelles commis à l'encontre de majeurs. d'information. De même, l'article 2 du projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, aggrave les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. C'est la proposition n° 15

des modifications apportées en commission des lois ont été guidées par la volonté de rendre plus efficace ce texte : nous ne voulons pas de mesures purement symboliques, au détriment non seulement des règles constitutionnelles, mais aussi de l'efficacité de la loi. Que retenir de l'examen en commission des lois ? La commission a d'abord adopté l'allongement à trente ans du délai de prescription pour les crimes sexuels et violents commis à l'encontre des mineurs. Elle a également adopté, sur l'initiative de François-Noël Buffet, une disposition innovante visant à faciliter le recours à l'obstacle de fait insurmontable, qui vise à suspendre la prescription. Elle a modifié le régime de prescription de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription. Concernant le harcèlement sexuel et moral, notamment commis sur internet, la commission a approuvé les modifications de l'Assemblée nationale en les enrichissant. Elle a ainsi adopté une disposition permettant de mieux lutter contre le cyberharcèlement en conférant de nouvelles obligations aux plateformes Concernant l'outrage sexiste, la commission des lois en a approuvé le principe tout en refondant le dispositif. En effet, elle n'a pas jugé opportun d'en faire une contravention : comme l'a rappelé le Conseil d'État au Gouvernement, la création d'une contravention relève du pouvoir réglementaire, et non du pouvoir Au regard de la gravité des faits et de la complexité des éléments constitutifs de l'infraction, qui devront être constatés par les policiers et gendarmes, la commission des lois a jugé plus pertinent d'en faire un délit. Néanmoins, afin de permettre une constatation en flagrant délit et une sanction rapide, la commission des lois a prévu l'application de la procédure de l'amende forfaitaire en matière délictuelle pour cette infraction. Concernant la répression des viols, commis sur majeurs ou sur mineurs, la commission des lois a approuvé, en en améliorant la rédaction, l'extension de la définition du viol adoptée par l'Assemblée nationale aux actes de pénétration forcés, commis commis non pas sur la victime, mais sur l'auteur des faits, au détriment de la victime : il s'agit des fellations réalisées de force sur de jeunes mineurs, qui n'étaient jusqu'à présent pas considérées comme un viol. Concernant la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, le Gouvernement est revenu sur ses premières déclarations. Initialement en effet, il avait annoncé la création d'une présomption irréfragable de non-consentement attachée à un seuil d'âge pour les mineurs. Une telle annonce, un peu précipitée, se dispensait d'une réflexion sur les pratiques judiciaires ou d'une évaluation de l'arsenal pénal existant. À l'inverse, la commission des lois a choisi de prendre le temps de la réflexion avant d'annoncer une évolution de la loi par la création d'un groupe de travail pluraliste, elle a proposé son analyse des défaillances actuelles dans la répression des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. Pourquoi un arsenal pénal si vaste est-il aussi peu connu et mobilisé ? Pourquoi les crimes sexuels font-ils autant l'objet d'une correctionnalisation ? Ce n'est pas parce que la loi est incomplète, et la seule création de nouvelles dispositions de nature pénale n'y changerait rien. Évidemment, comme nous l'avions déjà souligné dans notre rapport d'information, le Conseil d'État a considéré que de telles dispositions paraissaient contraires à plusieurs dispositions constitutionnelles. Il a rappelé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel empêchait toute création de présomption irréfragable de culpabilité, surtout en matière criminelle. Or la création d'une infraction qui reviendrait à créer une présomption irréfragable de culpabilité pour tout majeur ayant une relation sexuelle avec un mineur de quinze ans porterait une atteinte disproportionnée au principe de la présomption d'innocence et aux droits de la défense. Comme l'a rappelé le Conseil d'État, la seule circonstance que l'auteur « ne pouvait ignorer l'âge de la victime » ne répond pas à l'exigence constitutionnelle relative à l'élément intentionnel en matière criminelle. En conséquence, le Gouvernement a renoncé à son projet initial pour proposer la création d'une disposition interprétative concernant la contrainte morale ou la surprise pour les viols commis sur les mineurs de moins de quinze ans et la création d'une circonstance aggravante pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas d'acte de pénétration sexuelle. La commission des lois a choisi de modifier la disposition interprétative. Elle a supprimé la circonstance aggravante pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas d'acte de pénétration sexuelle. En effet, une telle disposition crée une possibilité supplémentaire de requalification du viol en atteinte sexuelle et accroît donc le risque de correctionnalisation. Le viol reste un crime. Surtout, la commission des lois a choisi d'aller plus loin : elle a décidé de protéger tous les mineurs victimes de viols, pas seulement ceux de moins de quinze ans, pas seulement ceux de moins de treize ans. En conséquence, elle a proposé la création d'une présomption de contrainte qui inverse la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs, lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d'âge significative entre l'auteur et la victime mineure. Ce sera à l'agresseur de prouver qu'il n'y a pas eu contrainte Cette disposition, plus souple que l'instauration d'une présomption simple reposant sur un seuil d'âge des victimes, permet de s'adapter à la diversité des situations et, surtout, de protéger tous les mineurs. Il convient de faire très attention à toute modification de la loi pénale : nous ne pouvons instrumentaliser son évolution au profit d'une communication politique Nous ne pouvons pas non plus simplifier de manière excessive le code pénal au risque d'affaiblir la protection actuelle des mineurs ! À cet égard, la commission des lois a également supprimé tous les « neutrons législatifs Enfin, la commission des lois a réparé les oublis du projet de loi. Ce texte ne parle en effet que de la réponse pénale. Or la prévention des violences est essentielle ! Cela doit être la priorité. C'est pourquoi elle a proposé que ce projet de loi porte véritablement les orientations de la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Je ferai miens les propos de Lamartine, qui a vécu en Saône-et-Loire : « J'ai eu le courage et le chagrin de vous déplaire, mais de vous déplaire pour vous servir. » Là, il s'agit de servir les victimes de violences sexuelles. bien ! La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, saisie pour avis.

je concentrerai mon propos sur les dispositions de l'article 2 qui ont plus particulièrement fait débat, dans un contexte marqué par la vive émotion causée par deux décisions judiciaires. Rappelons que nous partageons tous un même objectif, celui de mieux protéger les enfants contre les prédateurs sexuels, même si nous ne nous accordons pas nécessairement sur les moyens. L'objectif de la délégation est aussi de rendre impossibles de nouvelles affaires de Pontoise et de Meaux. Pourquoi ces affaires sont-elles survenues ? Parce que la définition du viol repose sur des critères- violence, menace, contrainte, surprise -qui font une large place à l'appréciation subjective du magistrat ou du juré. ces critères conduisent immanquablement à juger le comportement de la victime. Cette mise en cause d'une responsabilité supposée de la victime est d'ailleurs propre au viol : on ne reprocherait pas à quelqu'un qui s'est fait voler sa voiture d'en avoir une Quand il s'agit de victimes adultes, ces questionnements sont déjà très perturbants et injustes. Quand il s'agit d'enfants, ils sont inadmissibles, car ils conduisent à s'interroger sur leur prétendu consentement. Comment imaginer qu'un enfant puisse consentir à une pénétration sexuelle par un adulte ? Au terme de ses travaux, la délégation a acquis une conviction : les critères du viol ne sont tout simplement pas pertinents quand il s'agit d'enfants. La seule solution protectrice est d'instaurer dans le code pénal un seuil d'âge en deçà duquel toute relation sexuelle avec pénétration entre un adulte et un mineur serait un crime, sanctionné à la hauteur de sa gravité. Les critères de menace, violence, contrainte ou surprise n'entreraient plus en ligne de compte, et le consentement de la victime ne serait plus évoqué. La délégation a fixé ce seuil à treize plutôt qu'à quinze ans. Cet âge nous a semblé la limite universellement admise de l'enfance. De plus, nous avons souhaité séparer le débat législatif du débat moral quand on envisage un seuil de quinze ans, on en vient implicitement à un débat sur l'âge auquel on peut admettre que des jeunes aient une vie sexuelle. Or ce n'est pas le rôle du législateur. Nous avons eu aussi comme préoccupation d'éviter des plaintes contre un jeune majeur qui aurait des relations sexuelles avec un adolescent plus jeune. En ce qui concerne les droits de la défense, nous avons considéré que le seuil de treize ans garantit un écart d'âge suffisant entre victime et agresseur et que ce dernier pourra démontrer qu'il ne pouvait connaître l'âge de la personne avec laquelle il a eu un rapport sexuel. Nous ne sommes pas convaincus de l'inconstitutionnalité supposée de notre proposition, qui nous a régulièrement été opposée. Notre proposition est confortée par des spécialistes éminents. Dans une tribune récente, ils « réclament avec force la création d'un crime formel de violences sexuelles à enfants quand un adulte a une relation avec une personne mineure de moins de treize ans ». C'est très exactement ce que propose la délégation Le texte dont nous débattons répond-il à nos exigences ?

En effet, la notion de contrainte morale, dans l'appréciation du viol, laisse une part trop grande à la subjectivité. Pour nous, se référer à une différence d'âge « significative » entre victime et agresseur ou à l'incapacité de discernement du mineur n'empêchera pas le débat sur le consentement de l'enfant. Cette mesure n'empêcherait donc pas de nouvelles affaires du type de celle de Pontoise. Pour conclure, la solution que nous défendons nous semble être la plus protectrice des jeunes victimes. Combien de scandales faudra-t-il encore avant que le législateur ne crée une une nouvelle infraction réprimant le crime de violence sexuelle commis sur un enfant ? Mes chers collègues, au moment de l'examen de l'article 2, je vous demanderai de bien avoir à l'esprit l'enjeu de votre vote les dispositions proposées permettront-elles réellement de protéger nos enfants contre les prédateurs sexuels et de garantir une condamnation des agresseurs à la hauteur de la gravité des faits ? La parole

« Il n'y a pas de secrétariat d'État aux miracles » disait Françoise Giroud un an après la création du secrétariat d'État à la condition féminine en 1974. en 1974. En la matière, le temps est nécessaire, et nécessairement long. La domination masculine résiste parce qu'elle est universelle. Elle constitue, avec la prohibition de l'inceste, le point commun à toutes les cultures, à toutes les sociétés, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque. Pour Françoise Héritier, cette hiérarchie entre les sexes résulte d'une construction culturelle et ne correspondait pas initialement à une réalité biologique. Les hommes se sont approprié le corps de la femme pour mieux maîtriser la fécondité. On aurait ainsi longtemps accepté que le corps des femmes appartienne aux hommes et que les femmes soient les seules responsables du désir qu'elles suscitent, au point que cette soumission en serait devenue « paradoxale », selon le terme employé par Bourdieu. paradoxale parce que la domination masculine s'exprimant par une violence douce, insidieuse, elle a été intégrée par les femmes elles-mêmes. Les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent quotidiennement sont si ordinaires que les femmes s'y résignent,

le texte affirme le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre de mineurs et instaure ainsi une forme d'imprescriptibilité.

L'instauration d'une présomption de contrainte en deçà de treize ans créerait une zone grise en termes de répression pénale, laquelle pourrait inciter à se reposer exclusivement sur la qualification pénale d'atteinte sexuelle et donc mobiliser insuffisamment la qualification pénale de viol. Or telle n'est pas notre intention. La création d'une telle présomption ferait aussi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l'existence d'une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de treize ans.

que plus de 80 % des petites filles mineures atteintes d'un trouble mental font l'objet avant leur majorité d'atteintes sexuelles graves, que 91 % des mineurs autistes, filles ou garçons, font l'objet des mêmes violences. Il n'y a plus lieu de polémiquer sur les moyens juridiques. Nous avons un très bon dispositif, adoptons-le Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, travail a été effectué jusqu'ici par les associations féministes et celles qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que par les délégations aux droits des femmes des des deux chambres du Parlement, le sentiment prévalant est toujours celui de la maltraitance des victimes et de l'impunité des agresseurs. Le texte qui nous est soumis d'apporter une réponse législative à ce qui est surtout un immense chantier social et sociétal à ses balbutiements ! Quoi que l'on puisse penser de ses dispositions, la première chose qui frappe, c'est son relatif manque d'envergure. Qui peut vraiment penser que quatre modifications législatives suffiront pour lutter efficacement contre

La réalité de notre société, qui méconnaît encore souvent la gravité, la fréquence et la prégnance des violences sexistes et sexuelles, devrait nous inciter à plus d'ambition. La parole féminine qui s'est exprimée ces derniers mois et les #MeToo et #BalanceTonPorc qui ont déferlé sur les réseaux sociaux sont venus nous rappeler que les violences sexistes et sexuelles s'exercent sur nos concitoyennes de manière massive, sans distinction de milieu social ou professionnel. Ce mouvement, souvent présenté comme une libération de la parole des femmes, nous interroge d'abord sur le silence qui l'a précédé et qui, quoi qu'on dise, s'impose toujours à l'immense majorité des victimes. Ces problématiques ne sont pas nouvelles. Elles ont d'ailleurs été évoquées ici même, en février 2017, lors d'un débat lancé sur mon initiative sur le thème : « Violences sexuelles : aider les victimes à parler ».

d'apporter des réponses à ces atteintes majeures à l'intégrité même du corps féminin. Cette histoire remonte à loin. Longtemps soumise à une domination masculine sans partage,

En témoignent entre autres l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, le peu de place que les femmes occupent en politique, dans les conseils d'administration, à la tête des entreprises, aux postes à responsabilité. Les exemples sont nombreux, jusqu'à la circulation de la parole féminine elle-même sans cesse interrompue, ici ... et là. Les violences sexistes et sexuelles découlent d'une perception globale, directe ou indirecte, de la femme comme objet plutôt que comme sujet, perception que nombre de femmes elles-mêmes ont fini par intérioriser. Leur silence face aux violences sexistes et sexuelles n'est pas étranger

plainte contre son agresseur. Ce chiffre est certes impressionnant, mais il ne peut être imputé à la seule faiblesse supposée de notre arsenal législatif. Ce silence est lié aussi à ce qu'il convient d'appeler la culture du viol, qui consiste à faire porter Pour démonter cette culture du viol, il est nécessaire de rappeler inlassablement qu'une victime de harcèlement ou d'agression sexuelle n'est jamais responsable de ce qu'elle subit Il est indispensable de développer l'information et la prévention dans les écoles, les universités, les administrations, les entreprises, pour que les citoyennes et les citoyens puissent appréhender clairement ce qui relève d'une infraction sexuelle, le repérer, y réagir et surtout le dénoncer. Si tout cela n'est pas accompagné d'une valorisation de la place de la femme dans la société, les efforts déployés pourraient se révéler vains. Éducation et manuels scolaires ont un rôle important à jouer en la matière en faisant évoluer leur contenu. On ne peut pas se dispenser non plus, pour les victimes osant parler, d'un véritable accompagnement au moment du dépôt de la plainte, puis tout au long de la procédure. De même, si la police et la justice ne sont pas dotées des moyens financiers et des formations nécessaires à cette mission, il est à craindre que tout cela ne soit qu'un coup d'épée dans l'eau. Toutes ces questions méritent débat. Nos divergences seront probablement nombreuses. Convenons toutefois toutes et tous que ce sujet doit

madame la ministre, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, notre République se doit de protéger tous les siens et tout particulièrement les plus faibles. Elle se doit de poser des interdits, de sanctionner les infractions, surtout les plus inacceptables, mais elle doit aussi et surtout les prévenir. Votre texte, madame la ministre, affiche cette ambition. Pour ma part, j'évoquerai tout particulièrement les violences sexuelles sur mineurs,

preuve indéniable de notre volonté commune sur toutes nos travées de mieux combattre les violences sexuelles. Je pense à l'allongement de la prescription à trente à l'aggravation des peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, à l'aggravation des peines en cas de non-assistance ou non-dénonciation d'actes de mauvais traitement, ou encore la meilleure répression du harcèlement en ligne. Un article cristallise toutefois les débats, l'article 2, sur lequel portera l'essentiel de mon propos. Cet article introduit dans la définition du viol une protection particulière pour les mineurs de quinze ans. Les notions de contrainte et de surprise, constitutives d'un viol, pourront « être caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». Cette disposition interprétative va dans le bon sens, et je m'en réjouis. Toutefois, la proposition de notre rapporteur est plus protectrice envers les mineurs- tous les mineurs -et plus sévère à l'encontre des accusés. elle inverse la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d'âge significative entre l'auteur et la victime mineure. Il appartiendrait donc, selon la proposition de notre rapporteur, à l'accusé de démontrer l'absence de contrainte. Cette présomption de contrainte permettrait d'assurer la protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, qu'ils aient douze ans ou qu'ils en aient seize, s'ils manquent de maturité ou de discernement. L'âge n'est pas synonyme de maturité ou de discernement. D'aucuns proposent d'instaurer un seuil d'âge à treize ans. Si la fixation d'un seuil peut être considérée comme un renforcement de la protection et la sacralisation d'un interdit sociétal, elle

Le juge pourra en effet considérer ce seuil comme une limite, ce qui pourrait l'inciter à privilégier la qualification d'atteinte sexuelle au détriment de la qualification pénale de viol.

Ne prenons-nous pas le risque d'assister à la même puissante incompréhension que celle qui a jailli lors de l'affaire dite « de Pontoise » ? Le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants ont d'ailleurs indiqué ne s'être jamais montrés très favorables à l'introduction d'un seuil d'âge dans la loi, en précisant qu'il convenait d'être extrêmement prudent sur toute disposition qui introduirait une certaine automaticité dans l'application de la loi pénale. Le Gouvernement a renoncé, après l'avis du Conseil d'État du 15 mars 2018, à instaurer un seuil, eu égard aux risques d'inconstitutionnalité, que notre rapporteur a parfaitement exposés, et sur lesquels je ne reviendrai pas.

équilibre fragile entre la nécessaire répression des infractions sexuelles, en particulier à l'encontre des mineurs, et le respect de la cohérence du droit pénal, de la conformité à la Constitution. Je salue son courage et la qualité de

en rapprochant la peine encourue en cas de viol et en cas d'atteinte sexuelle avec pénétration, est que les affaires de viols sur mineur dans lesquelles contrainte et surprise seraient compliquées à établir soient trop facilement requalifiées en délits d'atteinte sexuelle. Ainsi, ce qui était jugé hier comme un crime en cour d'assises pourrait être communément considéré demain comme un délit au tribunal correctionnel. Il faut avoir à l'esprit que, en moyenne, une procédure pour viol dure environ six ans tandis qu'une procédure pour agression sexuelle dure environ deux ans. Et qu'un jury populaire n'est pas une garantie de fermeté dans la sanction, loin de là. Aussi, pour certaines victimes, le choix d'accélérer le processus peut être libérateur. Pour d'autres, un viol jugé en correctionnelle serait plus difficile à surmonter, car elles n'auraient pas le sentiment

En effet, cela a été rappelé, 11 % des victimes de viols ou d'agressions sexuelles seulement portent plainte. La grande majorité des victimes n'a ni la force ni l'endurance d'engager des recours.

Nul ici ne sous-estime la complexité du sujet, mais nul ici ne peut nier que chacun de nous porte comme un devoir, une conviction, une volonté la protection farouche de tous les mineurs. Aussi, sur un tel sujet, il appartiendra à chacun, en son âme et conscience, mais avec raison et discernement, de se prononcer. La parole

suffisent pas à effacer les points contestables, et ils sont nombreux. Vous avez ainsi renoncé à instaurer un seuil d'âge minimum en dessous duquel toute relation sexuelle d'un mineur avec une personne majeure est interdite, pour des raisons que vous avez tenté d'expliquer tout à l'heure et sur lesquelles nous reviendrons évidemment au cours du débat, réduisant ainsi

madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, qu'elles concernent les mineurs ou les majeurs, qu'elles se déroulent sur internet ou dans la rue, toutes les violences sexuelles et sexistes doivent être dénoncées et combattues avec fermeté. Pour cela, il apparaît nécessaire de mieux sensibiliser et éduquer l'ensemble de la société à cette problématique qui connaît un développement croissant. Aussi, nul ne saurait remettre en question, au sein de cet hémicycle, les objectifs poursuivis par ce projet de loi. loi. Sur un sujet complexe, on ne peut pas apporter une réponse hâtive. Il y va de la qualité de la loi. Je me félicite donc que la commission des lois de notre assemblée, dans sa sagesse, ait pris le temps de la réflexion avec la création d'un groupe de travail pluraliste sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. Car il apparaît clairement que, si ce projet de loi contient des évolutions importantes du code pénal, son effectivité et sa clarté nécessitent en revanche des améliorations. Ainsi, la commission des lois a notamment réparé des oublis majeurs du projet de loi en le complétant par des volets relatifs à la prévention des violences sexuelles et sexistes et à l'accompagnement des victimes, déjà prévus par le Sénat lors de l'adoption, au mois de mars 2018, de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Afin de faciliter les poursuites criminelles en matière de viol commis à l'encontre de mineurs, la commission des lois a choisi de protéger tous les mineurs, sans distinction d'âge, en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d'âge significative entre l'auteur et la victime mineure. La commission a également prévu de transformer la contravention d'outrage sexiste en un délit,

destiné à préserver les personnes importantes ou, au contraire, vulnérables, telles que les enfants, par la transmission de règles morales implicites assimilées inconsciemment par les individus. Si l'inceste figure parmi ces interdits universels, force est de constater que la seule existence de ce tabou n'est pas suffisante pour empêcher la transgression de cet interdit. Dans nos sociétés contemporaines, différentes lois pénales ont donc explicité ces interdits et ont progressivement protégé les mineurs des violences sexuelles dont ils peuvent être les victimes. Les différentes auditions menées par notre groupe de travail, piloté par notre collègue Marie Mercier, ont permis de souligner la nécessité de parler de ces violences particulières et de l'importance de les faire sortir de la zone d'ombre où le tabou les maintient parfois. C'est pourquoi, de façon générale, nous nous félicitons de toutes les occasions données au législateur d'évoquer les violences sexuelles commises sur mineurs, dans l'espoir que les débats tenus dans cet hémicycle servent de caisse de résonance et participent à la prévention de ces actes, que nous appelons de tous nos voeux. Je voudrais à ce titre rappeler, parmi les constats dressés par notre rapporteur, l'aspect éludé par ce projet de loi que sont les violences sexuelles exercées par des mineurs sur d'autres mineurs. Comme le montre une étude, à Paris, 44 % des mis en cause pour un viol commis sur un mineur sont également mineurs et, parmi eux, 42 % avaient entre dix et quatorze ans au moment des faits. Ces quelques données montrent, me semble-t-il, l'importance que nous devons porter à l'éducation préventive auprès des plus jeunes quant au respect du corps d'autrui, et la vigilance qui incombe aux adultes encadrant les mineurs au moment de la découverte de leur sexualité. Elles posent également la question de l'accompagnement des enfants coupables de telles violences sexuelles. Madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les interventions des uns et des autres montrent qu'il n'y a pas aujourd'hui d'opposition à l'objectif fixé par le deuxième titre de ce projet de loi. Cela devrait augurer de débats apaisés. Les seuls désaccords qui persistent concernent en réalité les modalités pénales de cette protection et la latitude accordée aux juridictions dans cette tâche. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur la pertinence de l'intégration des deux premiers titres du projet de loi à un texte également consacré à la lutte contre les violences sexistes, s'inscrivant, lui, dans le cadre de la politique du Gouvernement de promotion de l'égalité entre les sexes. Certains aspects de la réforme de la justice, qui sera examinée à l'automne, auraient mérité d'être discutés avec la question du risque de correctionnalisation lié à la création d'un délit d'atteinte sexuelle avec acte de pénétration- je pense à la création des tribunaux criminels. Sur l'allongement du délai de prescription de vingt à trente ans, je vous avais fait part de mon cheminement lors de l'examen de la proposition de loi, adoptée au Sénat le 27 mars dernier. Si cet allongement est acceptable dans une perspective protectrice à l'égard des victimes, en revanche, la transformation en une imprescriptibilité déséquilibrerait considérablement l'échelle des prescriptions, adossée à celle des peines. Concernant le coeur du projet de loi et la question de la fixation d'un seuil d'âge en dessous duquel une pénétration sexuelle commise par un majeur sur un mineur devrait être systématiquement regardée comme un viol, mon groupe est particulièrement partagé. La multiplication de seuils parallèles à celui déjà fixé par l'article 227-25 du code pénal relatif à l'atteinte sexuelle est de nature à créer des confusions. Les exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives à la présomption d'innocence ne facilitent pas la rédaction de cette disposition, en raison de l'impossibilité d'établir des présomptions en matière criminelle. D'un autre côté, il y a les arguments tout à fait compréhensibles des victimes mineures de violences sexuelles qui considèrent qu'une interdiction absolue aurait permis de mieux les protéger. Nous sommes donc majoritairement favorables à la rédaction équilibrée proposée par notre rapporteur, mais certains d'entre nous soutiendront la proposition d'établir un seuil à l'âge de treize ans. Il faut d'ailleurs souligner que ces deux dispositions ne sont pas contradictoires, mais complémentaires.

commis contre l'intégrité corporelle des mineurs de quinze ans, qui reprennent, là aussi, les travaux effectués par notre groupe de travail. Enfin, nous tâcherons de nous inspirer de l'héritage discret, mais décisif, de Simone Veil au moment d'évoquer la lutte contre les violences sexistes. S'inscrivant dans la même « maternité », ma collègue Françoise Laborde et les autres membres de la délégation aux droits des femmes ont formulé des propositions intéressantes visant à diversifier les outils de lutte contre les violences sexistes. Nous soutenons, bien entendu, les dispositions venant condamner les raids numériques. En revanche, si certains d'entre nous sont favorables à l'élargissement de la définition du harcèlement sexuel proposé par l'Assemblée nationale, d'autres craignent qu'elle ne vienne créer la confusion avec le délit d'outrage sexiste proposé à l'article 4, le risque étant, comme l'a souligné le Défenseur des droits, que l'on vienne « contraventionnaliser » le harcèlement sexuel par l'ajout des comportements à connotation sexiste à la définition du harcèlement. Nous soutenons les améliorations introduites par notre rapporteur sur ce point. Sur le nouvel outrage sexiste, si nous sommes en plein accord avec l'objectif de faire cesser ces comportements intolérables, nous sommes plus partagés sur les réponses à apporter à ces agissements. La réponse législative que nous apportons m'apparaît difficilement applicable, puisqu'elle repose en grande partie sur du flagrant délit. Pour conclure, le groupe du RDSE, fidèle à sa tradition, votera selon ses sensibilités et selon le sort réservé à ses amendements. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, madame la rapporteur, chère Marie, mes chers collègues, membre du bureau de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, c'est avec espoir et attention que j'ai étudié puis amendé ce projet de loi dont on ne peut qu'approuver les intentions, puisqu'il vise à lutter contre certaines violences sexuelles et sexistes. Je ne reviendrai pas longuement sur l'article 1 du projet de loi. Ses dispositions me paraissent adéquates et conformes aux attentes des victimes. En effet, l'allongement du délai de prescription pour les infractions sexuelles commises sur les mineurs participe d'une véritable reconnaissance de la difficulté pour une victime de ces agressions de les admettre et de porter plainte. Allonger à trente ans la durée de la prescription en la rendant identique à celle qui s'applique, entre autres, aux crimes de guerre démontre aux victimes l'importance accordée à leur souffrance.

La proposition de la commission des lois visant à créer une présomption de contrainte en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs mérite d'être examinée avec intérêt, car elle introduit la notion d'incapacité de discernement du mineur et la différence d'âge significative. Cela laisse entendre également que c'est à la personne majeure de faire preuve de discernement. Cette disposition est primordiale et a toute mon approbation, car elle permet de protéger les victimes mineures, toutes les victimes mineures sans seuil d'âge. En ce qui concerne la création d'une contravention pour outrage sexiste, je note que le texte lui accorde une véritable place dans notre code pénal, ce que le projet de loi initial ne s'était pas résolu à déterminer. Peut-être les violences dont sont victimes les femmes et parfois les hommes dans la rue, les transports en commun, au travail, à la maison, cesseront-elles enfin d'être considérées comme anecdotiques. Il est important, ne serait-ce que d'un point de vue moral, de leur accorder une véritable considération. Cette infraction permettra de faire prendre conscience aux auteurs de la gravité de l'agression dont ils se rendent coupables, et ce serait déjà un bon début. Pour que la dissuasion soit effective, je suis favorable à la transformation de la contravention en délit. Cependant, je doute que la création de cette infraction soit réellement dissuasive ou que le paiement d'une amende et, éventuellement, l'accomplissement d'un stage soient suffisants pour empêcher la récidive. Il me semble plutôt que, pour ce qui est des insultes, des sifflets, des moqueries, il est avant tout question d'éducation et de prévention. Nous devons avoir à coeur de protéger les victimes d'agressions sexuelles ainsi que les victimes de sexisme, j'y suis particulièrement sensible et je sais que, dans cet hémicycle, nous le sommes tous. Vous l'aurez compris, j'ai tout de même un certain nombre de réserves à émettre sur ce texte, et la première d'entre elles est son manque d'ambition sur un point essentiel.

J'avais formé à cet égard beaucoup d'espoirs. Peut-être le Gouvernement compte-t-il agir en ce sens dans les prochains mois ? Nous l'espérons. Si tel est le cas, vous pourrez compter sur l'engagement et la détermination des sénatrices et des sénateurs de cet hémicycle pour répondre aux questions que soulève ce sujet majeur. La parole

L'examen des articles nous permettra de nous exprimer sur les autres aspects du projet de loi. Il y a quelques mois, le grand public découvrait un angle mort dans la protection des enfants contre les violences sexuelles, un angle mort que les spécialistes connaissaient, je le précise, afin de lever les suspicions de ceux qui pensent que nous légiférons sous la pression des faits divers ou des médias. Cet angle mort se résume ainsi : en l'absence de violence, menace, contrainte ou surprise, la qualification de viol ne peut être retenue à l'occasion d'une relation sexuelle avec pénétration d'un majeur sur un enfant, et c'est la qualification d'atteinte sexuelle sur mineur qui est retenue. Cette qualification délictuelle est jugée en correctionnelle ; elle n'est pas criminelle et n'est donc pas jugée en cour d'assises. Or je considère, et nous sommes nombreux à partager ce point de vue, qu'une relation sexuelle avec pénétration entre un majeur et un mineur doit être un crime et non un délit, qu'il est indispensable qu'un seuil d'âge, en l'occurrence treize ans, soit fixé et qu'il ne saurait être question ni de maturité sexuelle ni de discernement d'un enfant qui consentirait à un acte sexuel avec un adulte. Lorsque nous parlerons de l'outrage sexiste, vous nous direz probablement, madame la ministre, que cette contravention a une vertu éducative et qu'elle pose un interdit clair et lisible. Si ce raisonnement, que je partage, est fondé pour l'outrage sexiste, il l'est,, pour le crime de violences sexuelles sur enfant. Depuis l'automne dernier, nous avons tous, à un moment ou à un autre, été d'accord, le Président de la République, les délégations aux droits des femmes du Sénat et de l'Assemblée nationale, vous-même, les experts, les professionnels, les associations, les magistrats, je pense particulièrement au procureur Molins, Molins, pour fixer un seuil dit de non-consentement et punir comme un viol une relation sexuelle entre mineur et majeur. Or, où en sommes-nous aujourd'hui ? Cette volonté a été torpillée à la fois par le Conseil d'État et par la commission des lois de notre assemblée. Deux arguments ont tourné en boucle : l'inconstitutionnalité pour cause d'irréfragabilité d'une prétendue présomption et l'absence de l'intentionnalité de l'auteur. l'inconstitutionnalité n'est, à mon sens, pas sérieux. D'une part, la rédaction soumise au Conseil d'État n'est pas celle que nous vous proposons aujourd'hui. Nous nous étions fourvoyés sur la voie de l'extension du viol. Nous suivons aujourd'hui une tout autre logique. On ne pourra donc pas opposer l'avis du Conseil d'État à l'amendement que nous vous soumettons.

Et je cite à cet égard Jean-Marc Sauvé qui soulignait, à l'occasion d'un colloque de droit constitutionnel : « Sous le ciel de la Constitution, plusieurs analyses [ ...] peuvent donc coexister, même si, cela va de soi, le Conseil constitutionnel a le dernier mot. Les arbitrages rendus par le Gouvernement n'ont pas pris en compte la subtilité du droit constitutionnel et ont donné au Conseil d'État le premier et le dernier mot. En ce qui concerne l'exigence d'une intention qui, comme le disait Aristote, fait la culpabilité et le délit, je ne vois pas en quoi la création d'un crime de violences sexuelles sur enfant y porterait atteinte. Il n'y a pas de pénétration involontaire, alors qu'il y a, en effet, des homicides involontaires. Je ne vois pas davantage comment un pénis peut se trouver involontairement dans l'anus, le vagin ou la bouche d'un enfant. En revanche, j'ai bien identifié un argument qui revient chez ceux qui combattent ce crime de violences sexuelles : la crainte de traîner aux assises un auteur qui ne serait pas coupable, car il serait la victime d'une Lolita.

En bref, alors qu'on devrait légiférer pour mieux protéger les enfants, on légifère en réalité dans le souci de protéger des auteurs de pénétrations sur enfants ... C'est inadmissible ! ... au motif qu'ils auraient « ignoré » qu'ils pénétraient un enfant. des sceaux, madame la secrétaire d'État, dans cette affaire, le droit constitutionnel et les principes généraux du droit pénal sont dévoyés. Ils ne sont que les alibis de la résistance d'une minorité active de notre société à poursuivre devant les assises les prédateurs auteurs de violences sexuelles sur enfants. J'ai noté que le Gouvernement n'a pas déposé d'amendement rétablissant les alinéas 14 et 15 de l'article 2. Vous avez même annoncé que vous retiriez cette infraction d'atteinte sexuelle avec pénétration, c'est bien. bien. Dès lors, que reste-t-il de cet article ? Une aggravation des peines et des dispositions interprétatives. Tant mieux, mais nous sommes loin des ambitions annoncées. Entre le dépôt du projet de loi, la lecture à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, la société s'est mobilisée.

À cette fin, il propose d'allonger certains délais de prescription, de mieux sanctionner les viols commis à l'encontre des mineurs, de mieux réprimer les faits de harcèlement sexuel ou moral, notamment lorsqu'ils sont commis en ligne, et de verbaliser les outrages sexistes. Le groupe Les Indépendants souscrit pleinement aux objectifs fixés par ce texte. Nul ici ne peut en contester la légitimité, car nous sommes tous convaincus de la nécessité de donner un coup d'arrêt à un certain nombre de violences qui continuent à se produire, allant parfois jusqu'à l'inhumain. Trop souvent et en trop grand nombre, les mineurs demeurent victimes d'infractions sexuelles ou, plus largement, de violences à caractère sexuel.

et, d'autre part, d'une proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Ces deux contributions furent le fruit d'un groupe de travail, dont j'ai fait partie, mis en place en octobre 2017. Toutefois, je voudrais vous faire part d'un certain nombre de remarques. En premier lieu, comme je l'avais déjà évoqué non seulement en commission, mais également à cette tribune, j'aurais souhaité, à titre personnel, que la notion d'imprescriptibilité figurât à l'article 1. reste persuadé, permettrait que la parole des victimes soit enfin libérée. En deuxième lieu, je regrette que le Gouvernement ait fait le choix de la procédure accélérée. Sur une question aussi grave et complexe, qui engage l'avenir de notre société à travers nos enfants, il eût été préférable de laisser le temps du débat au Parlement. En troisième lieu, je déplore que le Gouvernement n'ait pas associé le Sénat à l'élaboration de ce projet de loi, alors que, précisément, la commission des lois avait constitué un groupe de travail pluraliste sur ce sujet. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants partage la même ambition que le Gouvernement. Il votera donc en faveur de ce texte, dont l'effectivité et la clarté ont été améliorées par la commission des lois du Sénat. La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Madame la présidente,

Plus que jamais, notre action doit être guidée par l'article 1 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, proposée par Olympe de Gouges à l'Assemblée nationale en 1791. C'est dans cet esprit, je le sais, que notre collègue Marie Mercier a travaillé avec responsabilité et détermination sur ce projet de loi, afin de le renforcer et d'en faire un véritable outil au service des femmes et des jeunes filles de France en particulier. Je tiens à lui témoigner mon total soutien et ma reconnaissance pour la tâche qu'elle a su accomplir, parfois dans des conditions difficiles, mais jusqu'au bout, sans jamais abandonner. Merci, chère collègue Aujourd'hui, il est urgent d'agir pour lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes. Au premier trimestre de 2018, les services de police ont traité environ 170 affaires par jour. Sur ces trois mois, le nombre des viols a augmenté de 12 %. La montée des violences envers les femmes doit nous alarmer, tant le respect de leur intégrité physique et psychologique est devenu un véritable enjeu de société. Ces violences peuvent frapper chacun d'entre nous, au sein de notre environnement, de nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, et touchent, il faut le rappeler, toutes les catégories sociales. Un crime Un crime sexuel n'est pas seulement une abomination. Il constitue aussi un violent et profond traumatisme chez sa victime, parfois jeune. Comment accepter plus longtemps que la prescription intervienne au bout de vingt ans ? Vingt années ne suffisent pas toujours pour purger la peur et refermer les plaies. Il est donc indispensable de porter ce délai à trente Au sein de la commission des lois, il nous a d'ailleurs paru nécessaire d'empêcher la prescription de courir avant que la victime puisse elle-même dénoncer les faits aux autorités. Nous devons aider les victimes à libérer leur parole, afin qu'elles puissent engager des poursuites pénales pouvant aboutir à des résultats concrets. Bien évidemment, notre collègue Marie Mercier a été particulièrement attentive à la question des viols commis sur les mineurs, crimes particulièrement monstrueux qui traumatisent à jamais de jeunes enfants ou de jeunes adultes en construction. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a validé sa proposition de « présomption de contrainte » pour les actes sexuels les impliquant, déjà votée par le Sénat en mars dernier. Par ailleurs, il est grand temps de faire comprendre que les femmes ne sont pas des objets. En ce sens, la transformation de l'outrage sexiste en délit permettra de garantir aux femmes le respect de chacune d'entre elles sur la voie publique, à condition, bien évidemment, que davantage de moyens financiers et humains y soient consacrés. Mes chers collègues sénateurs et sénatrices, soyons unis pour combattre tout ce que les femmes subissent dans certaines villes et dans certains quartiers, des pressions, aussi psychologiques que physiques, qui les contraignent à accepter l'enfermement et qui les placent sous la dépendance masculine, allant même parfois jusqu'à les rendre invisibles. Il n'a jamais été aussi urgent d'envoyer un signal clair et fort à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, pour qu'elles sachent que la loi et la République sont à leur côté et ne les abandonneront jamais, afin de les protéger et de préserver

beaucoup d'entre vous le savent, j'ai consacré une part importante de ma vie publique à la protection de l'enfance, comme ministre en charge notamment de la famille et comme président de conseil départemental. J'ai ainsi eu l'honneur de défendre devant le Parlement, en 2007, la loi refondant la protection de l'enfance, adoptée à l'unanimité des deux chambres. Puisque Mme la secrétaire d'État et plusieurs d'entre vous, chers collègues, nous ont invités à être dignes de l'héritage de Simone Veil, je m'efforcerai, moi aussi, d'être à la hauteur de la fidélité que je lui dois, ayant été l'un de ses plus proches collaborateurs- je pense être le seul dans ce cas au sein de notre assemblée. Je n'ai qu'un objectif aujourd'hui, protéger les enfants et, plus précisément, protéger tous les enfants, et pas seulement une partie d'entre eux. Et je pense que la solution proposée par la commission des lois est la plus protectrice de toutes. Je veux rappeler que le droit pénal français est déjà un droit très protecteur de l'enfant victime, même si nous pouvons bien sûr encore l'améliorer, en particulier sur la prescription et sur la caractérisation de la contrainte qui entre dans la définition du viol ; j'y reviendrai. Aujourd'hui, le viol d'un enfant, c'est vingt ans de prison ; l'agression sexuelle d'un enfant, dix ans ; l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, Fort heureusement, les magistrats sont généralement d'une grande sévérité pour réprimer ces crimes et ces délits graves. C'est d'ailleurs le moins que l'on puisse attendre face à l'intolérable. Nous proposons d'aller encore plus loin. Il peut, certes, y avoir des décisions de justice choquantes. Mais le meilleur moyen de corriger les erreurs d'une justice qui reste une oeuvre humaine n'est pas de modifier la loi pénale quand elle est déjà sévère, c'est de rénover et de réformer la justice, comme le Sénat l'a proposé depuis plusieurs années, et de la réformer vigoureusement. Si nous devions modifier la loi pénale chaque fois que le réquisitoire d'un procureur ou le jugement d'un tribunal nous choque, alors nous ferions fausse route et nous serions, de surcroît, inefficaces. Dans un État de droit, la régulation du fonctionnement des tribunaux se fait par l'appel et la cassation. À la suite d'un avis très rigoureux du Conseil d'État, le Gouvernement a dû renoncer à créer une présomption irréfragable de culpabilité, c'est-à-dire une présomption qui ne permet pas à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence, pour tout acte sexuel avec pénétration commis par une personne majeure sur une personne mineure de quinze ans. L'Assemblée nationale l'a suivi. En effet, nos droits fondamentaux prévoient, et c'est à notre honneur, que même le pire des assassins a le droit de plaider sa cause et de tenter de démontrer son innocence pour se disculper. Un tel principe ne saurait connaître de dérogation et n'en a jamais connu dans notre République. Il n'en connaît d'ailleurs nulle part en Europe. Tout automatisme dans la sanction d'un crime est un déni de justice. Le rôle du juge consiste à réunir les preuves du crime et à apprécier la réalité de l'intention criminelle. La présomption irréfragable de culpabilité ferait de lui une sorte de greffier, voire de robot, constatant des faits sans avoir de responsabilité d'appréciation pour les qualifier ou non de crimes. Dans des affaires si graves, il faut pourtant entendre chacun, respecter les droits de la défense de l'accusé et vérifier la réalité du crime avant d'enfermer pour vingt ans un individu. C'est parce que cette fonction aura été bien remplie que la peine sera légitime, si lourde soit-elle, et nous souhaitons bien sûr qu'elle soit lourde quand la victime est un enfant. Ces principes ont une force considérable. Le Gouvernement l'a admis, comprenant qu'il ne suffisait pas de bonnes intentions pour faire de bonnes lois. Il a donc inventé une formule consistant à éclairer la cour d'assises sur l'interprétation de la notion de contrainte morale, qui permet de définir un viol sans violence ni menace. nettement meilleure que la précédente, mais elle comporte deux faiblesses : d'une part, l'introduction d'un seuil d'âge, quel qu'il soit, ne permet pas de protéger tous les enfants ; d'autre part, c'est une simple disposition interprétative, sans portée juridique, qui aurait pu relever en réalité d'une instruction de la Chancellerie aux procureurs. La solution adoptée par notre assemblée le 27 mars dernier, à l'unanimité moins trois voix, me paraît bien meilleure, car elle est plus sévère pour l'agresseur. Aujourd'hui, l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que le procureur de la République ait prouvé sa culpabilité. Notre solution consiste à énoncer une présomption simple de contrainte morale quand le discernement de la jeune victime, quel que soit son âge, rend impossible un consentement libre et éclairé. Cette présomption de viol imposerait à l'agresseur de prouver son innocence, sa culpabilité étant présumée jusqu'à preuve contraire. Il y aurait donc bien une inversion de la charge de la preuve. La différence d'âge entre l'agresseur et la victime serait également prise en compte. Un agresseur de trente ans ne pourrait jamais se prévaloir de l'éventuel discernement d'une victime de douze ans pour s'exonérer de son crime. Cette solution est beaucoup plus rigoureuse pour l'accusé et beaucoup plus protectrice pour la victime que la proposition actuelle du Gouvernement. Certains de nos collègues, qui ont pourtant voté la proposition de loi adoptée par le Sénat en mars dernier, ont considéré qu'il fallait en réalité reprendre la proposition initiale du Gouvernement, en décidant que « constitue un crime puni de vingt ans de prison, tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant de moins de treize Mes chers collègues, je vous invite à être cohérents par rapport au vote de mars. La mise en oeuvre d'une telle proposition apporterait aux enfants une fausse protection : comment pourrait-on justifier que la protection d'un enfant de « treize ans moins un jour » soit différente de celle d'un enfant de « treize ans plus un jour » prenne soudain un caractère criminel, simplement parce que l'aîné des deux aura fêté son dix-huitième anniversaire ? Que décideront les juges en cas d'agression sexuelle sur des enfants de treize à quinze ans si le législateur marque lui-même la nécessité de différencier ces victimes au regard de la loi pénale ? Nous avons bien sûr à nous préoccuper de la constitutionnalité de ce que nous votons, car, la Constitution, ce sont les droits fondamentaux des Français. C'est ainsi que nous continuerons à mériter d'être considérés comme la chambre de la réflexion, de la sagesse, des libertés, mais aussi comme une assemblée réellement protectrice de l'enfance en danger.

en ce qui concerne non seulement la protection de l'enfance, mais aussi, plus largement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est précisément parce que notre droit est déjà fourni en la matière que le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui est court. C'est aussi parce que la loi est déjà dense que nous entendons travailler sur ce qui,

J'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer à cet égard. Le projet de loi que nous portons, avec Nicole Belloubet, vise à renforcer la condamnation des violences sexistes et sexuelles. C'est vraiment l'objet de ce texte. Il n'y a pas de volets préventifs, parce que ces derniers soit sont déjà dans la loi, soit relèvent de politiques publiques et pas du législatif. S'ils sont absents du projet de loi, cela ne veut pas dire qu'ils soient absents de l'action du Gouvernement. Je pense notamment à la mise en oeuvre de lois déjà existantes. Vous le savez toutes et tous, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la loi prévoit que l'éducation à la vie affective et sexuelle dans le monde éducatif. Cette loi n'est pas mise en oeuvre. Nous avons travaillé, avec Jean-Michel Blanquer, sur un audit depuis maintenant plusieurs mois, mené auprès des établissements et des rectorats, qui nous a révélé ce que nous pressentions déjà et qui nous était remonté par les acteurs de terrain, à savoir que cette loi n'est pas mise en oeuvre. Nous avons donc lancé une circulaire à l'adresse des recteurs, demandant à chacun de faire appliquer cette loi, qui prévoit trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par année scolaire. Nous leur avons aussi adressé un catalogue mentionnant l'ensemble des associations qui ont un agrément pour intervenir en milieu scolaire. Nous avons par ailleurs relancé une tournée d'interpellations auprès des associations, afin que ces séances puissent être mises en oeuvre et menées réellement par des personnes compétentes et spécialistes. En outre,

sexistes et sexuelles. Avec la mallette des parents, nous communiquerons avec les parents sur ces questions de manière très claire. Vous le voyez, il y a une volonté, de la part de mon collègue Jean-Michel Blanquer et de la mienne, d'agir pour l'éducation face aux violences sexistes et sexuelles, même si la question ne relève pas du présent projet de loi. De la même manière, vous avez appelé notre attention sur les dispositions concernant l'égalité salariale. Par définition, celles-ci ne figurent pas dans un texte qui vise à mieux condamner les violences sexistes et sexuelles. Néanmoins, nous avons pris un certain nombre de dispositions importantes, qui ont été, il est vrai, très peu relayées dans les médias, et je le déplore, dans le cadre du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

de calculer et de publier les écarts de salaires. C'est un pas important vers la transparence des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Ces employeurs disposeront alors de trois ans pour résorber ces écarts de salaires ; passé ce délai, ils s'exposeront à des pénalités financières. Ce sont des dispositions très importantes. Cela fait plusieurs générations

de telles inégalités. Ce sont des dispositions législatives. Je vous fais grâce des dispositions des politiques publiques, afin que nous ayons le temps d'entrer dans le coeur des débats, mais je suis bien sûr à la disposition de toute sénatrice ou de tout sénateur qui souhaiterait que nous puissions évoquer ce sujet en parallèle.

qui a permis de faire progresser la France sur les questions touchant à la place des femmes dans la gouvernance des entreprises. On dit, en Corse, que c'est à la fin de la cueillette que l'on compte les figues. Il est donc un peu tôt, six mois après le lancement de la grande cause du quinquennat, pour faire un bilan de celle-ci, puisque, comme son nom l'indique, elle est quinquennale. Je propose que nous fassions le bilan et le droit d'inventaire à la fin du quinquennat.

de lutte contre les violences conjugales, mis en place, dans chaque département, sur notre initiative, autour des préfets. Il y aura un partage d'informations entre la police, la justice, les travailleurs sociaux, les élus locaux, afin de mieux repérer, en amont, les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales et de pouvoir les écarter du domicile conjugal.

d'interpeller les témoins. Nous avons conscience du rôle clé joué par les témoins de violences sexistes et sexuelles, qu'il s'agisse de violences intrafamiliales ou de harcèlement de rue. C'est un combat culturel que nous devons mener. J'évoquerai également le plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les universités,

la mention d'un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans. Bien sûr, cela pourrait avoir le mérite de la clarté, de la simplicité et je comprends que vous puissiez faire cette proposition. Si nous ne l'avons pas retenue, c'est pour un certain nombre de raisons. La première s'attache à la dissociation

s'attache au fait qu'il pourrait paraître difficile de créer une infraction purement formelle en matière criminelle, c'est-à-dire sans prise en compte de l'élément intentionnel. J'ai bien entendu ce que vous avez indiqué de manière extrêmement concrète, mais il n'empêche qu'il semble toujours important d'apprécier la réalité de l'intention criminelle, pour reprendre un propos du

s'appliquer aux faits qui ont déjà été commis, puisque, vous le savez, il y a un principe à valeur constitutionnelle intangible de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère. Je ne vois pas très bien comment on pourrait pallier cette difficulté. La force de la disposition

Vous évoquez en outre, madame Gatel, la nécessité de renforcer les moyens de la justice. J'aurai l'occasion d'y revenir, ils seront effectivement renforcés, jamais assez, certes, mais en tout cas de manière extrêmement volontariste par le gouvernement actuel : plus de 1,6 milliard d'euros, 6 500 emplois, etc.

et au Conseil d'État, les distinguant bien l'un et l'autre, en revanche, je suis vraiment en désaccord profond avec la phrase que vous avez prononcée quand vous avez énoncé que le Gouvernement avait le souci de protéger les auteurs des violences à enfants.

n'est évidemment pas la volonté du Gouvernement, je voulais juste le rappeler devant vous. Monsieur le président Bas, je dois vous rendre hommage pour ce que vous avez le courage de dire quand vous énoncez que, dans un État de droit, la régulation des cours et des tribunaux se fait d'abord par

La discussion générale est close. J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination et du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence sont parvenues à un accord. la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie n'est pas parvenue à un accord. Nous reprenons l'examen du projet de loi,

le caractère transversal et obligatoire de la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui relève à la fois de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le diagnostic a été posé par différentes autorités

dans cet amendement : la prévention, bien sûr, la condamnation des agresseurs, mais aussi l'accompagnement des victimes. C'est pour cela qu'il nous a paru important que, en tête de ce texte, figurent cette ambition et ce principe de travail pour plus d'efficacité.

transversal et obligatoire de la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les moyens à y consacrer. Vous savez que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, je l'ai détaillée auparavant, est une priorité

texte est l'un des piliers d'un dispositif global et cohérent, dans le cadre de la grande cause nationale du quinquennat annoncée par le Président de la République. Je ne reviendrai pas sur les dispositions que j'ai déjà citées. Le fait que le secrétariat d'État dont j'ai la charge soit rattaché au Premier ministre garantit ce travail interministériel et le caractère transversal de la lutte nécessaire contre les violences sexistes et sexuelles, qui est la première priorité de cette grande cause du quinquennat. Le fait que nous défendions conjointement ce projet de loi, avec la garde des Sceaux, en est une illustration parmi d'autres que j'ai mentionnées

exécuté, pour avoir un budget sincère, par opposition au précédent budget, jugé insincère par la Cour des comptes. Ce sont 420 millions d'euros qui sont mobilisés en interministériel par l'ensemble du Gouvernement.

J'en profite pour préciser que, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, il n'y a aucune baisse des subventions versées aux associations nationales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Certaines ont même été augmentées : par exemple, le Collectif féministe contre le viol recevra 60 000 euros supplémentaires pour l'année qui vient.

pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail dans l'ensemble des régions de France, afin de couvrir et de mailler véritablement le territoire. Il s'agit de faire en sorte que ces politiques publiques ne soient pas

comme je l'évoquais voilà quelques instants. À ce titre, nous rappelons que ce texte est l'une des pierres angulaires de l'engagement pris par le Président de la République de faire de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles le début de sa grande cause nationale du quinquennat. Mais ce n'est pas, bien sûr, l'alpha et l'oméga de cette grande cause du quinquennat, c'est l'un des piliers d'un édifice que nous commençons, ensemble, à bâtir. Le 25 novembre dernier, le Président de la République, lorsqu'il a décrété la grande cause du quinquennat, a également présenté un plan d'action

mesures interministérielles importantes ont été présentées. Les mesures élaborées en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations patronales pour faire reculer les violences sexistes la diffusion de la culture de l'égalité à l'école, je n'y reviens pas, sur les grands plans de formation initiale et continue des forces de l'ordre, des personnels soignants, des magistrats, des enseignants, conformément aux objectifs de la circulaire de mars dernier, sur le lancement de la plateforme de signalement en ligne gérée par les forces de l'ordre pour informer et orienter les victimes de violences sexistes et sexuelles, et sur l'ouverture, d'ici à la fin de l'année, à titre expérimental, de dix centres de soins de psychotraumatismes pour les victimes de violences.

c'est le contraire qui aurait été surprenant ! Toutefois, dans notre démocratie, il me semble essentiel, au sujet d'une politique aussi importante pour la prévention des souffrances endurées par des personnes vulnérables, que vous puissiez vous adosser à un débat ayant lieu au sein de la représentation nationale. Pour cela, l'instrument adéquat, c'est la loi d'orientation et de programmation. Il ne suffit pas

à maintenir le caractère de loi d'orientation et de programmation que nous avions déjà donné à notre proposition de loi au mois de mars dernier.

pour que les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des enfants diminuent mécaniquement. En amont, tout le travail de prévention, d'accompagnement des victimes, de mobilisation des services de police, de formation de la justice exige d'autres

mobilisation interministérielle. Car, voyez-vous, le Parlement n'est pas simplement une encombrante institution par laquelle il faut passer régulièrement, c'est aussi une force et un point d'appui pour les ministres quand ils réalisent des grandes choses. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

n'inversons pas les rôles, nous avons déposé des amendements, et nous souhaitons qu'ils soient approuvés. J'ai cru comprendre que la commission préférerait qu'ils soient intégrés dans l'annexe. Ce n'est pas notre demande.

La France a ratifié le 4 juillet 2014 la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. L'obligation de créer un nombre suffisant de centres d'hébergement fait partie des engagements de la convention. En France, 400 000 femmes ont été victimes de violences conjugales, physiques et/ou sexuelles, au cours des deux dernières années, selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales parue en 2016. La faiblesse des ressources de certaines femmes, l'absence de réseau de solidarité familiale ou amicale et la difficulté à trouver rapidement des logements adaptés constituent souvent des obstacles majeurs à la volonté des femmes d'échapper aux violences dont elles sont victimes, au sein du couple, marié ou non, mais également en risque de mariage forcé ou bien encore victimes d'autres violences telles que l'esclavage domestique ou la traite des êtres humains. La stratégie de l'agresseur est souvent d'isoler ces femmes victimes de leurs familles et de leurs amis. L'offre d'hébergement dédiée aux femmes victimes de violences et les possibilités de relogement qui leur sont offertes sont des clés indispensables dans le parcours de sortie des violences conjugales selon le site du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant, ces places restent insuffisantes. Afin d'aider toutes les femmes victimes, l'augmentation des places d'hébergement devra se poursuivre et se renforcer pour répondre aux besoins.

l'avis du Gouvernement ? Madame la sénatrice, votre engagement est connu de longue date sur cette question de la défense des femmes victimes de violences. Je partage bien évidemment l'intégralité du constat que vous avez formulé,

à préciser que l'ensemble du Gouvernement est mobilisé pour l'hébergement des femmes victimes de violences et pour les mettre à l'abri. C'est l'un des axes prioritaires de la lutte contre les violences et pour la protection des femmes et des enfants. Ce sera l'un des objectifs majeurs des contrats locaux contre les violences conjugales que j'évoquais tout à l'heure, qui seront conclus auprès de chaque préfet, dans chaque département, au plus près de la réalité de chaque territoire. J'ajoute que nous avons annoncé en comité interministériel, le 8 mars dernier, la garantie de 5 000 nouvelles places d'hébergement pour les femmes victimes de violences et

des places qui sont disponibles. Nous sommes donc en train de travailler à cette plateforme de géolocalisation, qui sera accessible aux travailleurs sociaux, à la police, à la justice, aux élus locaux et qui permettra de savoir en temps réel le nombre de places disponibles dans tel centre d'hébergement. L'objectif est de pouvoir mettre au plus tôt

Outre que ces financements reposent exclusivement sur l'impôt local, les départements, ils créent une situation très inique, car ils dépendent de la volonté politique de tel ou tel pouvoir local. Je ne comprends donc pas que vous ne puissiez pas suivre cet amendement.

Le scrutin est ouvert.

dès 2017 par la mission de consensus coprésidée par Flavie Flament et le magistrat Jacques Calmettes et réunie à la demande de notre collègue Laurence Rossignol, alors ministre chargée des droits des femmes. Ces travaux ont largement contribué à faire évoluer les positions et à déverrouiller les blocages qui existaient. Cette évolution n'allait pas de soi il y a encore quelques mois : souvenons-nous des débats au cours de l'examen de la loi dite Fenech-Tourret sur la réforme de la prescription en matière pénale ! Il s'agit bien évidemment d'une avancée attendue par les victimes, en particulier pour celles qui, en raison de leur âge ou de leurs liens familiaux avec l'auteur des agressions, ont été incapables de révéler sur le moment les violences subies. les victimes sont parfois atteintes d'une amnésie traumatique qui les empêche de parler. Nous nous devions de prendre en compte, dans la loi, ces situations dramatiques pour permettre aux personnes concernées d'engager une procédure judiciaire, mais aussi pour mieux sanctionner les auteurs de viol et prévenir la récidive.

Ne fermons pas la porte à une telle évolution et laissons la réflexion se poursuivre. Peut-être y arrivera-t-on aussi ! Pour l'heure, la délégation soutient l'article 1, qui va dans le sens des recommandations qu'elle a formulées dans ses travaux récents sur les violences faites aux femmes. La parole

Benbassa, sur l'article. Le Parlement a été saisi à plusieurs reprises ces dernières années de textes relatifs à la prescription, celle des crimes commis sur les mineurs, bien sûr, mais aussi le régime général de la prescription en matière pénale, qui a été réformé en 2017. J'ai été mobilisée sur ces textes, qui sont parfois guidés par l'émotion légitime suscitée par l'impunité dont bénéficient encore bien trop d'auteurs de violences sexuelles. Forte de ce travail et des rencontres que j'ai pu faire avec différents acteurs, tant associatifs que judiciaires, je dois dire que ma position a évolué sur la question particulière des violences sexuelles subies par les enfants. Bien sûr, on pourra allonger la prescription jusqu'à la faire disparaître, cela ne garantira jamais à une victime qui parle vingt ou trente ans après les faits d'obtenir justice. Il faut faire preuve d'honnêteté en la matière : que restera-t-il après un temps si long ? Quelle enquête digne de ce nom pourra être menée ? Et que ressentira la victime, qui aura enfin pu parler et qui verra son agresseur relaxé faute d'éléments suffisants ? Ces questions, il me semble qu'il est de notre responsabilité de ne pas les éluder. Nous ne devons pas faire croire aux victimes que l'allongement de la prescription serait un remède miracle. L'accompagnement des personnes qui parlent très longtemps après les faits me paraît être particulièrement important, et ce tout au long de la procédure. Il faut recueillir leurs plaintes dans de bonnes conditions, mais surtout les préparer à ce que la vérité judiciaire, dictée par les principes de l'État de droit, contredise la vérité intime de ce qu'elles ont vécu.

Je soutiendrai donc l'allongement de la prescription proposé par l'article 1, tout en étant convaincue que la priorité, qui doit être celle de tous, est d'aider les victimes à parler plus tôt. C'est à cette condition que nous serons véritablement à leurs côtés.

à compter de la majorité de la victime, je reste convaincue qu'il ne faut pas fixer de limite à l'action publique à l'égard de ces crimes. Du point de vue des victimes, ce couperet n'est pas compréhensible. Je persiste donc dans cette conviction

en effet de publier un sondage, qui révèle que 70 % des Françaises et des Français sont favorables à l'imprescriptibilité du viol, quand il est commis sur un mineur. Je tiens aussi à rappeler un chiffre 37 % des victimes de violences sexuelles lorsqu'elles étaient mineures ont subi des amnésies traumatiques qui ont duré jusqu'à quarante

imprescriptibles. Avec tout le respect dû aux victimes de ces atrocités, ne peut-on pas établir une analogie avec les violences sexuelles sur les enfants ? Ces enfants devenus adultes n'ont-ils pas le droit, aussi, d'être reconnus comme victimes plusieurs années après les faits ? Je comprends les arguments expliquant que les preuves seront difficiles à apporter et que cela sera peut-être vécu comme une double peine par les victimes. Mais laissons-leur au moins la possibilité d'engager les poursuites ! Aujourd'hui, 16 % des femmes et 5 % des hommes déclarent avoir subi des viols ou tentatives de viols au cours de leur vie. Les chiffres sont de plus en plus terrifiants et, si les violences subies pendant l'enfance meurtrissent, les violences sexuelles détruisent plus encore. La victime est surexposée à d'autres violences et elle peut développer des comportements à risque contre elle-même et contre la société. Si la victime n'est pas réparée, elle peut souffrir de ce de violence tout au long de sa vie.

La qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte aux plus faibles de ses membres et la femme blessée dans son corps en fait partie. Les violences faites aux femmes touchent aux droits fondamentaux que sont l'égalité et la dignité. Elles doivent faire l'objet d'une attention particulière, aussi bien dans la prise en charge des victimes que sur le plan de la prévention et de la répression de ces actes. Le législateur doit garder en ligne de mire que son seul objectif est de protéger les femmes et les enfants de toutes les violences sexuelles. Le Sénat- je m'en réjouis -a fait évoluer le projet de loi, de telle sorte que soit notamment ajouté un volet relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes et à l'accompagnement des victimes.

en affirmant le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs, par le biais

Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d'État,

Cette situation remet en cause la capacité effective de ces victimes à déposer plainte dans les délais de prescription définis par la loi. C'est pour cette raison que je propose à notre Haute Assemblée de reporter le point le point de départ du délai de prescription en cas de constat par un médecin de l'existence d'une amnésie post-traumatique. Madame la secrétaire d'État, le 15 mai 2018, vous répondiez à mon collègue député Philippe Dunoyer qu'un tel amendement reviendrait à inscrire dans le code pénal une prescription indéterminée. Il n'en est rien ! Cet amendement reviendrait à inscrire dans le code pénal un délai de prescription de trente ans, qui serait effectif à partir de la majorité des victimes

nous pouvons inscrire cette disposition dans la loi.

Certains nous opposent l'incapacité de pouvoir apporter des preuves, le moment venu. D'autres nous disent que le droit à l'oubli est nécessaire et qu'il existe un problème constitutionnel,

et il faut souvent attendre que sa situation soit stabilisée pour qu'elle puisse enfin parler et que les procédures puissent être engagées.

la prescription des crimes commis sur les mineurs, en permettant, dans certains cas, un allongement très significatif de cette prescription. Il prend en compte la situation des personnes qui commettent des crimes de façon répétée sur les mineurs. Il prévoit

nous estimons qu'une telle mesure serait inconstitutionnelle. J'ajoute que cet amendement ne revient pas à rouvrir des prescriptions déjà acquises. C'est ce qui fait que l'amendement que nous vous proposons ne soulève, du point de vue du Gouvernement, aucun problème de nature constitutionnelle. Par ailleurs, cet amendement étend la prescription de trente ans aux crimes de violences sur mineur ayant entraîné une mutilation. Cela permet notamment d'incriminer, et donc de réprimer, l'excision. est également étendue aux crimes de meurtre ou d'assassinat commis sur un mineur. Toutefois, dans un souci de cohérence et de lisibilité de notre droit, ces ajouts ne sont pas insérés à l'article 7 du code de procédure pénale, comme le proposait l'Assemblée nationale, mais dans l'article 706-47 qui vise toutes les infractions sexuelles et auquel renvoie cet article. Je crois que cet amendement répond à des objectifs qui sont partagés

Pourquoi seuls les crimes contre l'humanité sont-ils imprescriptibles ? Parce que le nombre massif de victimes et l'ampleur des actes réprimés permettent facilement, même des dizaines d'années après les faits, de procéder à des condamnations sans erreur possible,

Quel alibi pourrait-il évoquer ? La prescription a pour objectif d'empêcher les erreurs judiciaires, en interdisant que des procès ne se tiennent dans des conditions empêchant le bon exercice des droits de la défense.

plus difficile à supporter pour la victime. Enfin, je rappelle que, depuis une décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a souligné qu'« aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit l'imprescriptibilité pour les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale », ce qui semble réserver l'imprescriptibilité aux seuls crimes graves affectant l'ensemble de la communauté internationale. De surcroît, il serait contraire au principe d'égalité devant la loi pénale de prévoir l'imprescriptibilité pour certains crimes de droit commun, tout en continuant à prévoir un régime de prescription pour d'autres délits encourant les mêmes peines. On ne pourra envisager l'imprescriptibilité des crimes sexuels que le jour où la France renoncera à l'idée de prescription pour toutes ces infractions. Or il semble que la prescription ait, encore aujourd'hui, toute sa pertinence, notamment pour éviter des erreurs judiciaires et des mises en cause tardives.

C'est un arrachement brutal d'une partie de soi. C'est ensuite la sidération dans un mélange de dégoût, de honte, de faute et de peur. C'est l'absence à soi-même qui s'installe sans l'avoir commandée, un effacement, comme un instinct de survie. Un enfant violé ne parle pas, il ne le peut pas, il est empêché, parce que l'infamie vient d'un adulte, souvent d'un proche. Pour l'enfant, c'est la nausée, née du trouble et de l'outrage ultime. L'enfant, s'il est très jeune, ne pleure même pas, il n'est nul besoin de lui faire peur, il ne parlera pas, il n'a pas les mots, il ne sait pas dire. D'ailleurs, où, quand et à qui parlerait-il ? Puis, le mécanisme d'oubli se met en place, consciemment ou non. Comme je l'ai dit, l'enfant est amputé à jamais. Sa vie ne sera pas ce qu'elle aurait dû être.

l'enfant violé l'est pour toujours ! Dès le début, l'enfant a appris à vivre avec et met en place des stratégies d'évitement, de déni, de refoulement. C'est la réponse irrationnelle au choc initial, et cela tout au long de sa vie. Comment survivre, sinon ? Parler est si difficile, il y a quelque chose de honteux à le dire, à l'évoquer, à ce que les autres vont imaginer. C'est vous dans des images choquantes et c'est terriblement gênant. Si les parents ne sont pas les violeurs, c'est comme une barrière infranchissable. Comment le leur dire ? Alors on attend, on oublie. Et puis cela revient toujours et encore et, à la faveur d'événements particuliers, déclencheurs, on commence à s'exprimer et à parler. Alors oui, il faut du temps, beaucoup de temps parfois. à toutes celles et tous ceux qui, enfants, furent victimes de violences sexuelles le temps de se sentir prêts à porter plainte, parce que c'est justice ! Nous nous devons de permettre cela. Notre société si civilisée se doit de protéger les enfants, en envoyant un signal fort : les pervers- il s'agit bien de cela, n'est-ce pas ? -doivent pouvoir être poursuivis sans limite de temps grâce à l'imprescriptibilité. La parole L'histoire a son poids, elle a été, un moment, suivie par le droit, mais le temps passe

ceux qui sont touchés de la manière la plus violente qui puisse exister. C'est la raison pour laquelle je défends ce principe. Madame la garde des sceaux, je ne partage pas votre point de vue.

à l'allongement des délais de prescription étaient tellement vigoureuses et solides qu'elles ont, à l'époque, contraint les associations de victimes à attendre une meilleure occasion.

et d'autres, comme moi, s'abstiendront.

Je sais que la proposition du Gouvernement est une piste intéressante, car la pluralité de victimes dans le temps est une donnée que nous connaissons, permettant parfois que les auteurs soient confondus et, donc, condamnés. nous donnerons un avis favorable à l'amendement du Gouvernement et au sous-amendement de la commission, qui l'enrichit et l'améliore. S'agissant du reste, en tant que juriste, et puisque nous sommes ici pour faire la loi,

au constat suivant : pour qu'un crime soit jugé, un coupable condamné, dans un temps qui est celui de l'infini, il faut amener la preuve de la culpabilité or, mes chers collègues, d'une manière qu'il convient d'appeler réaliste, comment peut-on imaginer laisser croire

de la preuve. C'est tout à fait net ! On fait en sorte que la victime n'ait plus à se justifier et puisse passer le reste de sa vie

par le même auteur contre d'autres mineurs. C'est là que je rejoins les arguments de notre collègue François-Noël Buffet : il y a quelque chose

sous-amendement de la commission des lois, je peux partager tous les témoignages particulièrement émouvants qui ont été

étions arrêtés sur l'idée que vingt ans à compter de la majorité, c'était déjà un bon pas. Je crains que nous ne donnions beaucoup d'illusions

Mais, je suis à peu près convaincu que toutes les victimes pour lesquelles les faits sont prescrits pourront témoigner aux assises, et qu'il en sera nécessairement tenu compte par le jury. Quoi qu'il en soit, je comprends bien le sens de votre amendement et je voudrais rassurer Mme Michelle Meunier : l'imprescriptibilité, on en prend le chemin

la priorité que les pouvoirs publics doivent donner, dans leur politique, à l'accueil, à l'information, à l'accompagnement des victimes, car ce n'est pas dans trente ans qu'il faut porter plainte, c'est aujourd'hui, demain ou, au plus tard, la semaine prochaine ! Il est absolument fondamental d'inciter au dépôt de plainte, de l'accélérer et d'accompagner la victime pour qu'elle puisse être accueillie dans de bonnes conditions. Ne laissons pas croire, parce que nous parlons de la prescription,

le délai de prescription serait rouvert. Il me semble que, bon an mal an, on arrive ainsi à un compromis satisfaisant, qui renforce les droits de la victime souffrant de l'amnésie post-traumatique et ne vient pas perturber la hiérarchie des crimes au regard des règles de la prescription.

Le scrutin est ouvert.

Il nous semble que le caractère continu de l'infraction instaurerait par voie de conséquence une forme d'imprescriptibilité. Nous vous proposons donc de supprimer ces deux alinéas, en cohérence avec nos précédents votes.

pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Introduit sur l'initiative de notre commission des lois, les alinéas 6 et 7 de l'article 1 entendent compléter ce dispositif en affirmant le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs, par le biais du report du point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin. Nous considérons que cette disposition reviendrait à introduire de nouveau une forme d'imprescriptibilité, ce qui ne nous paraît pas souhaitable, d'abord, en raison du principe de proportionnalité des peines, mais surtout pour des raisons de principe. Aujourd'hui, seuls les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide sont imprescriptibles. Mettre au même niveau l'infraction de non-dénonciation des agressions sexuelles semble pour le moins inopportun. Nous demandons en conséquence la suppression des alinéas 6 et 7. Il est tout de même très curieux que l'imprescriptibilité revienne sans arrêt dans nos débats. C'est vraiment un réel problème

est à Mme le rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la disposition adoptée par la commission des lois. Il s'agit de faire du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, privations et atteintes sexuelles commises à l'encontre d'un mineur ou d'une personne vulnérable un délit continu et non plus un délit instantané. Tant que l'infraction aura lieu, c'est-à-dire tant que la personne continue de ne pas informer des infractions en cours, la prescription ne commencera pas à courir. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie,

qui reprend l'article 6 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Mme Mercier proposait d'affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des privations, mauvais traitements et violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables. Le caractère continu de l'infraction permet une amélioration de la protection des victimes en reportant le point de départ du délai de prescription de l'action publique. Cependant, conditionner ce report à la cessation de tous les éléments constitutifs de l'infraction pourrait limiter le renforcement de la protection souhaitée par Mme la rapporteur à cause de la fragilité juridique de cette rédaction. En effet, certains éléments constitutifs de l'infraction ne peuvent cesser- je ne vous relis pas l'article du code pénal. Je ne vois pas pénal. Je ne vois pas comment la connaissance des faits, élément essentiel de cette infraction, pourrait cesser. L'objet de cet amendement et donc de proposer une rédaction qui reflète une traduction juridique plus fidèle et plus sûre.

Le Gouvernement s'était opposé à l'adoption de cette règle de prescription dérogatoire lors des débats à l'Assemblée nationale en faisant notamment observer que cette disposition lui paraissait sans portée juridique. Cet amendement est différent, car il ne traite pas de la prescription, mais il tend à réécrire l'article 434-3 du code pénal afin de faire de ce délit un délit continu tant que les mauvais traitements se poursuivent et en l'absence de toute dénonciation, le délit sera commis et la prescription ne commencera donc à courir qu'à la cessation des mauvais traitements. Si, actuellement, le délit de non-dénonciation de mauvais traitements est instantané, il est constitué chaque fois que se commettent des mauvais traitements ou des agressions et que la personne qui en a connaissance ne les signale pas. Lorsque les violences ou les agressions sont habituelles et répétées dans le temps, chaque fait nouveau crée une nouvelle obligation de dénoncer et, par conséquent, un nouveau délai de prescription, lequel est désormais de six ans. Il n'est donc peut-être pas indispensable d'en faire un délai continu. Cela étant, en cas de mauvais traitements sur un mineur, identifier de façon isolée chaque infraction commise sur la victime n'est pas toujours très simple. Dès lors, il me semble qu'ériger le délit de non-dénonciation en délit continu peut se justifier. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement donnera un avis de sagesse sur l'amendement de la commission.

veut que soient engagées des poursuites contre quelqu'un qui a été témoin de violences ou de mauvais traitements sans intervenir, le délai de prescription soit aligné sur le délai de prescription des mauvais traitements eux-mêmes, par exemple des violences sexuelles. En effet, il est assez logique que la victime

ou d'agressions sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables à partir de la majorité des victimes. Cet amendement manque de clarté. Il n'est pas possible de reporter le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime, sans autre précision, puisque le délit de non-dénonciation est un délit sans victime directe. Il ne faut pas confondre le délit de non-dénonciation avec les délits ou les crimes qui n'ont pas été dénoncés.

du délai de prescription pour l'auteur d'un délit court à compter de la cessation d'un crime commis par un autre. C'est assez innovant, mais c'est assez déconcertant. Si nous faisions courir

comment l'on peut affirmer que l'enfant victime de privations, de mauvais traitements, d'agressions ou d'atteintes sexuelles ne serait pas recevable à se constituer partie civile à

En effet, l'article 9-3 du code de procédure pénale prévoit que l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique est une cause de suspension de la prescription. Il est inutile de préciser dans l'article 708-48 du code de procédure pénale qu'une expertise peut être ordonnée pour vérifier l'existence d'un tel obstacle ; cette possibilité va de soi. Une telle disposition n'est pas normative. Au surplus, l'article 708-48 ne traite que des expertises diligentées dans des procédures qui portent sur des crimes ou délits de nature sexuelle ou violente commis contre les mineurs prévus à l'article 708-47. Or l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique peut se présenter dans n'importe quelle affaire. Il est dès lors injustifié de faire référence à cette hypothèse uniquement pour certaines procédures.

C'est une période pendant laquelle la victime est dans l'impossibilité absolue de pouvoir révéler ce qu'elle a vécu. Cette révélation interviendra à un moment indéterminé à la faveur d'un événement particulier que nous ne sommes pas capables de définir précisément. Au moment où cet événement intervient, la victime revit immédiatement l'ensemble du drame dont elle a été victime. a été victime. Ce que nous demandons, c'est que le juge saisi du procès puisse saisir les médecins compétents en la matière- un, deux ou trois, peu importe -pour se faire confirmer l'existence ou non de ce traumatisme,

Le scrutin est ouvert.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

Le scrutin est ouvert.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

de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d'ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d'infraction sexuelle. Comme l'a souligné Mme la rapporteur, Marie Mercier, « c'est déjà la pratique dans nombre de parquets, notamment à Paris

Il s'agit donc d'inscrire dans le code de procédure pénale une méthode d'investigation déjà existante, mais encore contingente selon les territoires et les politiques pénales menées par chaque procureur. Cet amendement ne crée pas un « effet » en sous-entendant « qu'il n'est pas possible de diligenter des enquêtes en cas de prescription », comme cela a pu être affirmé en commission des lois. Il ne prévoit pas qu'une victime de faits prescrits n'a plus le droit de porter plainte en dehors des infractions listées. Simplement, en matière d'infractions sexuelles, comme le recommande le rapport annexé au projet de loi, le fait de mener des investigations pour vérifier que l'agresseur n'a pas fait d'autres victimes est encouragé. Cet amendement participe donc à la lutte contre l'impunité des agresseurs sexuels.

en matière d'infractions sexuelles. Même si elle n'aboutit pas sur le plan pénal, l'ouverture d'une enquête peut avoir un caractère réparateur pour les victimes, quand elle leur permet d'entendre des aveux, voire de recevoir des excuses de la part de leur agresseur, dans un contexte où ce dernier ne peut pas être poursuivi en raison de la prescription de l'action publique. Elle permet aussi, dans certaines circonstances, de vérifier que l'auteur présumé des faits dénoncés n'a pas commis d'autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé. L'enjeu peut donc être également d'éviter l'impunité d'éventuels prédateurs sexuels. La parole

temps, non par le policier, mais par le procureur de la République, qui pourra ainsi décider, soit de classer la plainte sans suite, soit de la retenir puis de la classer s'il estime que les faits sont prescrits.

celui-ci prévoit que la commission de nouveaux crimes sera une cause d'interruption de la prescription des crimes les plus anciens. Il sera désormais indispensable d'enquêter sur les faits les plus anciens et apparemment prescrits, pour vérifier si leur prescription n'a pas été

madame la ministre,

En dépit d'un consensus indéniable sur la nécessité de protéger les enfants de toute forme de violence, notamment sexuelle, le présent article a suscité de nombreux et vifs débats. Poser un interdit clair et précis dans le droit en ce qui concerne les relations sexuelles entre un adulte et un enfant afin de mieux sanctionner les auteurs et de protéger davantage les victimes, telle était l'ambition initiale du texte.

qui impose la criminalisation de tous les types d'infractions à caractère sexuel perpétrées contre des enfants et qui dispose que les États membres doivent adopter des dispositions législatives spécifiques et prendre des mesures

Je rappelle qu'un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles. Dans 80 % des cas, l'auteur de l'infraction est une personne du cercle de confiance de la victime.

il relève de notre devoir de législateur de garantir dans la loi la protection pleine et entière des enfants. Toucher à un enfant

L'article 2 du projet de loi est celui qui fait le plus débat. Les récentes affaires judiciaires, évoquées par Maryvonne Blondin, les revendications des associations et représentants des victimes, le choix initial du Gouvernement témoignent de la nécessité d'une protection totale et absolue de nos enfants face aux violences sexuelles. C'est en ce sens, et après de nombreux travaux, que la délégation aux droits des femmes a décidé de proposer la création d'une nouvelle infraction : le crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de treize ans par un adulte. Cette proposition est-elle inconstitutionnelle ? Les juristes et magistrats que nous avons consultés ont répondu non. La nouvelle infraction proposée n'est pas irréfragable, puisque, comme pour le délit d'atteinte sexuelle, il n'y aurait pas d'automaticité de la culpabilité. En effet, l'accusé pourra toujours apporter la preuve qu'il ne connaissait pas l'âge de la victime. En matière d'intentionnalité, maintenant, la démonstration est simple, car, comme l'a rappelé Laurence Rossignol, le simple fait d'introduire son pénis dans l'orifice d'un enfant est clairement une action volontaire et intentionnelle, comme l'a conclu la Chambre des Lords au Royaume-Uni en 2008. De plus, nos voisins anglais et danois ont inscrit des articles similaires dans leur législation depuis maintenant plus de dix ans, sans que jamais une violation des droits fondamentaux ait été soulevée. Certains nous ont reproché la création d'une zone grise, entre treize et dix-huit ans. Au contraire ! Il s'agit d'une gradation dans la protection des mineurs : aggravation de la peine de viol pour les mineurs de moins de

Je vous invite, mes chers collègues, à voter la proposition de la délégation aux droits des femmes, car elle permet une protection totale de nos enfants contre les prédateurs sexuels. Agissons aujourd'hui ensemble et laissons à la sagesse du Conseil constitutionnel le soin d'arbitrer entre les attentes de notre société et notre Constitution

à une désillusion. Les faits graves jugés à Pontoise et à Meaux ont ému. La société attendait de nous que nous puissions mieux protéger ses enfants de onze ans, de treize ans, mais aussi, soyons-en certaines et certains, ses enfants de quinze ans, contre les atrocités de certains adultes. Nos concitoyens attendaient que la loi rappelle fortement et clairement que la société protège ces enfants des prédateurs sexuels. Ils attendaient que ceux-ci ne puissent échapper à l'accusation de crime. vos annonces de l'automne ont donc été positivement perçues. Nous allions éliminer l'idée du consentement d'un enfant aux relations sexuelles avec un adulte. Nous allions renforcer la criminalisation de ces actes, ce qui répondait aux préoccupations des victimes et des associations militant dans ce domaine. Trop souvent, en effet, ces associations ont dénoncé les insidieux procédés à l'oeuvre dans les méandres des commissariats et des tribunaux. De telles méthodes conduisaient parfois à la correctionnalisation de ces crimes, pour gagner du temps, pour que la défense coûte moins cher, pour éviter l'aléa du jury ... » Bref, pour de bien mauvaises raisons, en somme, les agresseurs arrivaient, eux, à échapper à la peine que les violences qu'ils avaient commises méritaient. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'un rendez-vous manqué. Au gré de l'avis du Conseil d'État, vous avez contorsionné vos ambitions, pourtant claires : vous avez adapté la notion de consentement, tant et si bien qu'elle est devenue floue et qu'elle est désormais soumise à l'interprétation des juges. Nous sommes, selon moi, assez loin de la grande loi que vous revendiquez. En matière de droits et de protection de l'enfant, il n'y a rien de plus efficace que la loi qui s'énonce aisément Personne n'a le droit de te faire du mal. Aucun adulte ne peut avoir une relation sexuelle avec toi, et, si tu te sens en danger, c'est le rôle de tous les adultes de te protéger. » C'est avec de telles dispositions que nous aurions pu engager un beau programme de sensibilisation, de pédagogie, avec les professionnels de l'enfance.

peut avoir séduit et provoqué un adulte, qu'il peut avoir donné un consentement. Nous affirmons que ce n'est pas possible : l'adulte est responsable est à Mme Laure Darcos, sur l'article. L'article 2 du projet de loi suscite bien des interrogations de la part des professionnels de l'enfance, des familles et des professionnels de santé ; à juste titre d'ailleurs, car le fait qu'un viol puisse être requalifié en délit d'atteinte sexuelle, alors même qu'il y a eu pénétration sexuelle, a soulevé l'indignation de nombre d'entre nous. Pouvons-nous envisager un seul instant qu'un mineur consente librement à des relations sexuelles avec un majeur, alors même qu'il n'a ni la maturité ni le discernement nécessaires pour accepter de tels actes ? Pouvons-nous faire comme si l'acte sexuel subi par un mineur était sans conséquence pour son équilibre psychique et physique ? La délégation aux droits des femmes a souhaité fixer à treize ans l'âge en deçà duquel un enfant ne peut consentir à un acte sexuel. Elle a ainsi créé une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur.

que la commission des lois a décidé, pour sa part, de protéger tous les mineurs, quel que soit leur âge, en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs, lorsque ceux-ci sont incapables de discernement, ou en cas de différence d'âge significative entre l'auteur et la victime mineure. Au-delà des débats de juristes, lesquels sont, bien entendu, nécessaires, je souhaite redire avec force qu'un enfant n'est pas un objet sexuel, que nous lui devons une protection absolue et que nous devons sanctionner avec une extrême fermeté ceux qui abusent de sa vulnérabilité, de sa fragilité et de sa crédulité.

On ne peut plus rester dans l'entre-deux sur de tels sujets. Il faut dire clairement qu'aucun enfant ne peut donner son consentement de façon éclairée à un acte sexuel ; il faut dire clairement qu'il est interdit, pour un adulte, de faire subir un acte sexuel, une pénétration à un enfant.

le Conseil constitutionnel ne pourra pas dire autre chose que cela. Nous devons voter ces dispositions. C'est un vote de civilisation, un vote historique. Il ne faut surtout pas commencer à se noyer dans des détails de seconde zone ; et, si ces détails existent, il est temps de les écarter

sur la réalité du droit applicable. Or, si l'on veut légiférer, il faut au moins que l'on sache quelle situation nous voulons changer. Premièrement, j'entends dire qu'il faut absolument interdire les relations sexuelles entre un adulte et un mineur. Mais cette interdiction figure déjà dans

si c'est une agression sexuelle, c'est dix ans ; si c'est une atteinte sexuelle, c'est cinq ans ; et des circonstances aggravantes peuvent augmenter un peu la peine. Deuxièmement, j'entends dire qu'il ne faut pas que le consentement de la victime puisse servir à épargner la condamnation de l'agresseur. Mes chers collègues, je vous rassure, notre code pénal ne prévoit pas que l'on prenne en considération le consentement de la victime. Vous ne le saviez peut-être pas : c'est pourtant le code pénal, tel qu'il s'applique dans notre pays, et ce, fort heureusement,

on se rend compte qu'il ne s'agit pas de refonder notre droit pénal, pour ce qui concerne les viols commis sur des mineurs par des adultes : il s'agit simplement de l'améliorer. Les fondations sont solides, elles sont justes. La justice fonctionne dans l'écrasante majorité des cas ; et, quand elle dysfonctionne, elle sait se corriger elle-même.

ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, [ ...], dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable », c'est-à-dire dès lors que l'accusé n'est pas condamné avant même le procès

non seulement les victimes, mais aussi les droits de la défense, parce que ces droits sont au coeur même de l'organisation de notre société et des principes fondamentaux que nous avons tous collègues, c'est la raison pour laquelle votre commission, qui est inspirée des mêmes sentiments que vous, qui veut aller dans la même direction, se heurtant à l'impossibilité de créer une présomption irréfragable, a décidé de créer une présomption simple. Au fond, nous ne sommes pas si éloignés les uns des autres : en vertu de la présomption simple, l'accusé

d'aller, et nous sommes efficaces. En effet, au-delà de toutes les questions de grands principes, que je rappelle, car je suis sûr que vous les approuvez, comme moi, et que, pour vous non plus, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas secondaire, nous avons

Tout cela n'est pas sérieux : je tiens à vous le dire ! On ne peut pas construire le droit pénal sur de bonnes intentions : on doit le construire sur une conscience claire des réalités du droit applicable, des réalités du fonctionnement de la justice et de la protection des droits de l'homme et du citoyen

Il n'y a pas non plus ceux qui s'attachent à défendre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ceux qui s'essuieraient les pieds dessus. Nous sommes tous attachés aux droits de la défense et à la Déclaration des droits de l'homme

Il me semble qu'il y a un malentendu entre nous : nous n'en sommes plus à essayer d'étendre la définition du viol pour créer des présomptions, irréfragables. Nous avons abandonné cette voie, dans laquelle nous avons été nombreux à nous fourvoyer au départ, pour revenir à une autre approche juridique, qui consiste simplement à qualifier de crime une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de treize ans.

d'entendre, non vos explications- je n'ai pas à vous les demander -, mais votre interprétation de ces termes, car je crains de comprendre. Effectivement, il y a peut-être des petites filles qui ne sont pas totalement claires

En l'espèce, il ne s'agit pas seulement d'un changement de degré, mais un peu de nature. D'où notre proposition : il s'agit de faire en sorte que des choses qu'on pouvait se représenter par le passé ne soient plus acceptables pour le futur.

Tel est le pas que nous vous demandons de franchir ce soir, ni plus, ni moins : aller vers autre chose, d'une autre façon,

sont conservées. Il s'agit d'ajouter un crime de violence sexuelle sur les enfants de douze ans et moins. ! Nous voulons renforcer notre arsenal pénal pour lutter contre toute forme de prédation sur les enfants de cet âge particulier. Je ne comprends pas

Nous avons imaginé, avec des juristes et des instances compétentes, un nouveau dispositif, qui renforce la protection des enfants de notre pays. Nous vous demandons d'intégrer

Comment voulez-vous vous reconstruire, reconstruire le milieu familial, lorsque vous savez qu'un viol serait considéré comme un délit, non comme un crime ?

Je voudrais juste vous rappeler ces deux principes : le consentement doit être absolu et le discernement ne peut pas avoir d'âge. Évidemment, un petit enfant n'est pas discerné. Mais, je vous le dis en tant que médecin, les enfants ont une sexualité, une sexualité qui est à eux

qu'une petite jeune fille de seize ans sache ce qu'elle fait et qu'une autre de quatorze ans et demi ne le sache pas ? Ce n'est pas cela, la réalité. La réalité, c'est une sorte de clair-obscur